Monsieur le président du Sénat, a pris acte de la démission, à compter du 26 du samedi 25 novembre à 0 heure de Madame Nadège Lefebvre sénatrice de l'Oise. d'État, ministre de l'Intérieur a fait connaître qu'en application de l'article 320 du code électoral, elle a été remplacé à compter du samedi 25 novembre à 0 heure par Monsieur Jérôme, pas cher, c'est Nater de loi je ne sais pas s'il est présent. N'est pas présent mais au nom du Sénat tout entier je vous lui souhaite la plus cordiale bienvenue. Alors la parole est à monsieur Michel Calvet pour une mise au point sur un vote. Oui, tout à fait, Monsieur le Président, mon collègue Jean-François Longeau, membre du groupe de l'Union centriste a souhaité rectifier son vote sur l'amendement 1 97 c'est l'amendement qui était relatif à la suppression à la suppression de la réforme de la taxe d'habitation, il a été comptés comme votant pour cet amendement, or il souhaité voter contre cet amendement. Donc acte et donner de votre mise au point, elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l'analyse politique du scrutin. La parole est à madame Nathalie Goulet pour un rappel au règlement. pour une autre fois avec un un attentat de plus de 230 victimes dans une mosquée, après les attentats contre les chrétiens d'Orient notre Sénat devrait s'associer au deuil des victimes et et de l'Égypte, et je souhaite que, conformément aux dispositions de l'article 29 de notre règlement nous puissions que cette session budgétaire sera finie inscrire un débat sur la sécurité au Moyen-Orient qui me semble plus que jamais précaire et et nécessaire, c'est la raison de ce rappel au règlement et je vous remercie de bien vouloir inscrire à l'ordre du jour de nos travaux, L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2018 adopté par l'Assemblée nationale dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement 159 tournant à rassurer un article additionnel après l'article 9. Monsieur Longeau n'est pas là son vote a été rectifiée mais il ne défend pas son amendement donc nous passons à l'amendement. les amendements identiques oui alors l'amendement 179 monsieur Calvet. Oui, Monsieur le Président, cet amendement concerne le recyclage des produits en fin de vie et il vise à instaurer une TG. Éric TGAP Hamon qui permettraient de de financer la mise en place de plans d'économie circulaire et des conception dans les 100 entreprises françaises, elle concernerait les taxes des entreprises mettant sur le marché plus de 10000 unités de vente par an et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un 1000000 d'euros, elle serait appliquée uniquement sur les gros producteurs de produits non recyclables, pour les inciter à se tourner vers l'économie circulaire qui est extrêmement importante, sans pénaliser les petites entreprises, avec cette mesure, c'est la cohérence complète de la politique française en matière de gestion des déchets d'économie circulaire qui est en jeu, sans elle, c'est une prime à ceux qui ne travaillent pas bien qui s'appliquerait sur des produits quand même de grande consommation, tels que les jouets, les ustensiles de cuisine, de vaisselle, les articles de sport de loisirs, les matériels de bricolage et de bureautique, les fournitures scolaires en cahier, etc, qui en général n'ont pas de 2ème vie, donc c'est pour inciter à l'économie, au développement de l'économie circulaire, Monsieur le Président. Merci dans la discussion commune : l'amendement 251 défendue par monsieur Bocquet. Oui, merci Monsieur le Président, milite, chers collègues, le présent amendement permet aux unité de valorisation énergétique de contribuer à l'atteinte de l'objectif fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte de multiplication par 5 de la quantité de chaleur et de froid renouvelable de récupération livré par les réseaux, chaleur et de froid à l'horizon 2030 de plus ainsi, conformément à la directive européenne cadre sur les déchets de 2008, cet amendement permet de respecter la hiérarchie des déchets en incitant et en favorisant la valorisation par rapport à l'élimination, en effet, la directive déchets précise que la valorisation ne peut pas être assimilé à de l'élimination ainsi: est-il logique que les installations, réalisant une valorisation énergétique soient exonérés de TGAP enfin la loi de transition énergétique donne une priorité forte à la valorisation des énergies fatal et de récupération pour rappel, la valorisation énergétique représente un 1000000 de tonnes d'équivalent pétrole ou une tranche nucléaire ou 2000 éoliennes soit à il est totalement légitime de les exonérer de TGAP afin de permettre un développement plus conséquents, par ailleurs, seuls 16 unités arrivent à valoriser des produits non recyclables, je vous remercie.

pas l'anticipation, me semble-t-il, aujourd'hui, parler de réseaux chaleur de valorisation énergétique, ça ça me semble être l'objet des amendements, suivant là nous parlons de quoi nous parlons d'un élargissement de la TGAP pour des déchets qui ne sont aujourd'hui pas couverts par une filière de recyclage, donc sans doute ça répond à cet objectif d'avoir une fiscalité J. que d'avoir une taxe en amont sur les produits non soumis à une insolite élargie du producteur bon néanmoins tels que ces rédigé à la forme, et 3 amendements qui vient d'être défendu, me paraissent celui Hassan difficultés la 1ère c'est la définition même du Champ d'application puisque c'est appliquerait à l'ensemble des produits générateurs de déchets qui ne sont pas couverts par les filières c'est avec certaines exceptions bien sur les produits alimentaires par exemple énergétique, il faut avoir la notion est pour le moins floue, même si on nous dit que la liste sera précisé par décret d'aucun problème d'abord sur le Champ même de cette nouvelle TAG appelé la 2ème difficulté c'est sur l'impact on a auquel chiffrage combien ça représente, qui est le coût pour le consommateur final qui, de toute façon TGAP, donc il faudrait pouvoir disposer d'éléments relatifs à l'impact et enfin celui d'agression, ça nous renvoie une petit peu au débat d'hier soir est-ce que la taxation et la meilleure voie son doute pas là l'unique voie en tous les cas, mais est-ce que c'est la meilleure voie pour contribuer à Athènes subjectif de 50 pourcent de réduction de la quantité des déchets d'ici 2025 il y a d'autres voies et notamment il faudrait sans doute peut-être déjà crée les filières avoir inspecté la rigidité des producteurs, voir des des systèmes normatifs semble interdiction avoir des normes sur la la l'obsolescence etc etc, donc la taxation n'est sans doute pas la seule voie pas forcément non plus la meilleure, et il faut déjà que les filières existent et se mettent en place, avant d'envisager de le redire encore la fiscalité parce que, au final, c'est quand même un élargissement de la fiscalité, donc avis défavorables pour l'ensemble de ses raisons. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le Ministre. Excellent argument auquel se range gouvernement avis défavorable. Avis défavorable Michèle Canet pour. Explications de vote. Oui, tout à fait, monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, mais effectivement j'entends bien les arguments. Monsieur le rapporteur général non simplement l'ensemble des filières de valorisation des déchets se sont mises en place avec la responsabilité des producteurs, c'est-à-dire la participation des producteurs à la mise en place de filières, sinon on ne peut pas développer le recyclage des produits, il me semble que ce il y a bien fonctionné pour un certain nombre de produits peut-être tout à fait élargie, y compris au produit de très grande consommation et que la méthode ainsi proposé est tout à fait légitime en tout cas, elle ne fait que s'inspirer de ce qui a déjà été mis en place, donc c'est pas une novation et en la matière, on sait bien que il vaut mieux qu'il y a la responsabilisation des producteurs plutôt que la taxation sur le budget général, qu'il y a bien d'autres dépenses à financer, qui a bien d'autres besoins, donc il faut que l'on aille vraiment vers ce qui sont concernés par les produits pour inciter à leur valorisation, c'est vraiment le sens de de de cet amendement et on ne pourra agir sur ces produits que le jour où effectivement il y aura l'obligation pour les producteurs d'y mettre des moyens et donc des facto les industries de valorisation pourront se développer, ceci étant, moi j'entends l'argument les arguments qui ont été évoqués par rapporteur général et donc je retire l'amendement. Donc l'amendement 179 est retiré les 2 autres sont maintenues. Maintenu le 251 et le 513 aussi maintenu,

Oui, Monsieur le Président, c'est encore un amendement qui vise à mettre en oeuvre les actions prévues par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, hein, qui vise à à multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid renouvelable et de récupération par les réseaux de saveurs de froid et de froid à l'horizon 2030 donc il importe de trouver des mesures qui permettent véritablement il d'y aboutir et donc cet abonnement vise à exonérer de de taxe générale sur les activités polluantes, un certain nombre d'acteurs, pour leur permettre un développement de de ces outils, Si l'amendement 164 n'est pas défendu l'amendement 256 Monsieur Bocquet. Donc il était défendu par anticipation tout-à-l'heure continue de mon manque de vigilance en ce samedi matin, merci. Merci donc l'avis de la Commission, monsieur rapporteur général. ce sous-amendement, là nous sommes dans une l'idée d'exempter de TGAP des installations d'incinération de déchets à valorisation énergétique, donc je je précise tout de suite pour la bonne compréhension de l'Assemblée, que c'est l'installation bénéficie déjà d'un tarif réduit sur les exonérer ce serait contraire à l'objectif d'éviter la valeur d'éviter la sidération et de favoriser au contraire la valorisation, donc ce sera un petit peu antinomique par rapport à qui subjectif que j'astiquer tout à l'heure de réduire la quantité déchets incinérés de valoriser au mieux, c'est pour ça qu'il y a un tarif réduit actuellement mais pas une exemption donc ce serait évidemment contraire et c'est la raison à ce négatif et c'est la raison pour laquelle la Commission défavorable. Merci, Monsieur le Ministre défavorable aussi. Donc, nous allons passer au vote sur les 2 amendements, soit 23 et 256. En discussion quoi identique avec 2 avis défavorables commission et gouvernement, qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, ils ne sont pas adoptées nous poursuivons avec 3 amendements identiques, le 163 n'est pas défendu le 180 toujours monsieur

donc actuellement on sait que la TGAP taxe un certain nombre d'acteurs, y compris les les plus vertueux et moi aussi et ici cet abonnement visant à développer le dispositif d'incitation par un volet incitatif afin de récompenser les collectivités, entreprises qui contribuent au développement de l'économie circulaire et sont de plus en plus nombreuses, il suit le même objectif que les mesures de fiscalité déchets qui ont déjà été annoncées par le gouvernement et qui vise à diviser par 2 le nombre de déchets mise en décharge encore comme je l'évoquais hier beaucoup trop nombreuses et au recyclage de 100 pour 100 et des plastiques voulue par le président de la République, il créera une réflexion de de taxe générale sur l'activité polluante pour le stockage et l'incinération des déchets pour les collectivités, entreprises performantes en terme de valorisation Man hier des déchets et les seuils concernant le les entreprises concernées les collectivités pourraient être établie par décret, voilà Monsieur le Président, cet amendement. Merci l'amendement 255 Monsieur Bocquet. Oui, Monsieur le Président merci actuellement la TGAP fonctionne un peu comme une taxe essentiellement punitive, cette idée a été évoquée hier dans nos débats qui pénalise les collectivités et les entreprises, responsable de la gestion des déchets, lorsqu'elles sont contraintes traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage une nouvelle augmentation de la TGAP, telle qu'elle fut annoncée par le président de la République, pendant la campagne électorale fonctionnerait donc de la même manière elle pénaliserait en 1er lieu les collectivités qui doivent déjà subir une augmentation de la TGAP, suite à la loi de finances rectificative et qui sont déjà lourdement taxés sur les activités de gestion des déchets, cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif cette fois afin de récompenser les collectivités et entreprises qui contribuent ainsi au développement de l'économie circulaire suivra donc le même objectif que les mesures de fiscalité déchets annoncé par le gouvernement et contribuerait à diviser par 2 les déchets mis en décharge et au recyclage de 100 pourcent de plastique, annoncé par le président de la République, il créerait une réflexion de TGAP sur le stockage ou sur l'incinération des déchets pour les collectivités et entreprises performantes en termes de valorisation matière des déchets, les et permettant de définir les entreprises et les collectivités performant pouvant bénéficier de cette réflexion serait établie par décret cette proposition a part ailleurs été étudiés et validés par des constitutionnalistes qui ont conclu à sa constitutionnalité, notamment au regard du principe d'égalité devant l'impôt, je vous remercie. Le ministre voudrait prendre sur l'aspect constitutionnel j'imagine parce qu'il était évoqué, moi je regarde simplement les aspects plus pratique parce qu'il y a des modifications substantielles qui sont apportées par ces amendements hauteur de la TGAP médication technique, la difficulté, c'est que la lecture de l'amendement ne permet pas très bien de comprendre quels sont les critères qui permettent d'une part, d'apprécier la performance en matière de valorisation des déchets, et par ailleurs qu'il ne paierait quels sont les critères qui permettent de calculer les taux de réflexion proposée, donc il y a des taux d'infection, comment sont-ils calculés comment la performance apprécier et, enfin, on peut noter qu'il y a des qui sont similaires entre les entreprises et les collectivités donc, donc il y a pas de précisions à cet égard, donc la lecture du DVD des amendements ne permet pas. Concrètement, de justifier les modifications que substantielles qui sont proposées, donc c'est inviter favorable. Merci monsieur le ministre pour la ville, les gouvernements. Oui, merci Monsieur le Président, indépendamment des arguments du rapporteur général je réponds attend, bloqué sur la constitutionnalité et Jesper juridique, il me semble surtout que vos amendements prévoit une rupture d'égalité entre les assujettis à la TGAP,

serait diminuée, la TGAP acquittés par les exploitants des installations de traitement des déchets, et non par les apporteurs eux-mêmes et non pas possible sans méconnaître le principe d'égalité, d'appliquer des taux différents, les exploitants à raison de la qualité de leurs clients, les apporteurs de déchets, donc nous avons une difficulté juridique qui consiste effectivement à accepter si nous votre sur votre amendement si votre assemblée d'opter une différenciation qui serait de nature et créent une rupture d'égalité entre l'assujetti de cette taxe.

ensuite le 364 Monsieur Capet. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, c'est un amendement qui vise à doter les EPCI et les régions, en charge de l'élaboration et de la mise en oeuvre des plans climat air énergie territoriaux des schémas régionaux de du climat, de l'air et de l'énergie ou des schémas régionaux d'aménagement et développement durable et d'égalité des territoires, des moyens financiers et d'élaborer ces documents de planification stratégique donc ce que ce que vous propose cet amendement, c'est que ces acteurs territoriaux perçoivent une dotation de 10 euros par habitant pour l'élaboration d'un PC à T. et de 5 euros par habitant pour l'élaboration d'un S R C A ou d'un S. R. A. de B. T. je vous précise que c'est un qui avait déjà été déposée qui avait été adopté à la fois par les sénateurs et par les députés en 2016, mais il avait été retiré sur abonnement gouvernementale en 2016 je vous précise enfin qu'il est issu d'un engagement commun d'amorce de la des CFD régions de France 2 France urbaine de l'Association française du Conseil des communes et des régions d'Europe, de l'Association des Petites Villes de France, de la Fédération nationale des agences d'urbanisme de la Fédération des agences locales de maîtrise de l'énergie et du climat et du réseau des agences régionales de l'énergie et de l'environnement, c'est vous dire si c'est un engagement commun. Merci, cher collègue, l'amendement 594 n'est pas défendu, nous passons à l'amendement sort 24 équipiers quater madame la barbe. Oui, je ne peux rien ajouter à ce qu'a dit mon collègue qui a pu juste pour préciser que cette amendement fait dans son objet, a le même but que l'amendement de monsieur 1000 un peu plus précis dans sa rédaction et tient compte de la spécificité de la région Île-de-France, dans laquelle on a à la fois un EPCI, à savoir la métropole du Grand Paris des territoires et la Ville de Paris et pour donner un enjeu financier de cette mesure, si un tiers des collectivités ayant l'obligation de mettre en oeuvre schéma environnementale bénéficier en 2018 de cette fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, cela représenterait un groupe global de 300 millions d'euros, a rapporté à l'augmentation de la taxe qui a été votée hier soir d'environ 2 milliards

c'est vrai que les subject de la loi sont ambitieux mais comme souvent, les collectivités se sont vu transférer des moyens sans les moyens correspondants, elles auront du mal à atteindre les objectifs qui risque de rester à l'état d'intention et notre collègue Ronan Dantec, le disait hier soir sans les collectivités locales qui peuvent agir dans les territoires sur la vie quotidienne des gens, nous n'arriverons pas à atteindre les objectifs fixés, donc, encore faut-il le vouloir et aider les collectivités locales, bénéficier aussi des mécanismes de fiscalité écologique.

Le suivant le 277 rectifier n'est pas soutenu, donc il tombe le 365 rectifier monsieur C'est un amendement de repli qui ne vise que la dotation 10 euros pour l'élaboration d'un PC a voté. Très bien, merci l'amendement 595 n'est pas défendu. L'amendement 67 c'est Monsieur Ruquier qui le défend. C'était quand même un précédent mais qui a pas été défendu sa vie à transférer une part du produit de la TIC BE aux collectivités territoriales, engagé dans la tradition énergétique donc pour Madame de 10 euros par habitant.

Merci pour tous ces replis. L'amendement 596 n'est pas défendue donc. Nous allons demander l'avis de la Commission, monsieur, rapporteur sur les amendements qui ont été défendus.

parfois c'est aux EPCI parfois c'est région d'un montant qui va parfois 5 euros à 10 euros, notamment celles qui sont engagées dans des données schéma régional, aménagement et développement durable ou dans des schémas régionaux climat-énergie il y a plusieurs difficultés tout d'abord, il y a un coût, tout ça est très sympathique ça un coup c'était dit par notre collègue à l'instant 300 millions d'euros, c'est-à-dire des collectivités

entre collectivités, certains de ces amendements sont contradictoires entre certains affectés ce quasiment aux MPCI d'autres régions, d'autres 2, donc on a une vraie, vraie difficulté, dit à l'instant, tout ça mériterait c'est pas pour évacuer le débat, mais devant la contradiction entre ces amendements et difficulté à trancher tout cela mériterait pour le coup, clairement d'être discuté à la place des conférences, des territoires où la on doit avoir, pour le coup, Colette qui arrivent et qui connaît ces questions au devrait dans lequel ces conférences du territoire on discuter des relations entre l'État et les collectivités, et singulièrement des questions énergétiques, de ce point de vue, donc ça nous paraît un petit peu prématuré en tout cas, et n'pas à cette heure, les éléments d'expertise suffisante pour trancher à la fois en terme de montant et de répartition toute donc avis défavorable sur l'ensemble du monde. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre pour l'avis du gouvernement. Merci Monsieur le président, comme le dit très bien rapporteur général d'abord effectivement tout cela a un coût, pourquoi pas d'ailleurs à condition effectivement que cela soit concertée, il me semble quand même très bien dit monsieur le rapporteur général que dans le cas de la conférence nationale des territoires et notamment le le secrétaire d'État, Sébastien Lecornu a déjà eu l'occasion, me semble-t-il, de vous dire qui était à l'écoute de toutes ces propositions de ce travail, mais aussi les travailleurs important de fait, le ministre d'État émises à la maison des territoires, il me semble que sur des montants aussi importants avec un mécanisme qui certes touche attentat universalité budgétaire mais qui a été fait auparavant, notamment je pense de TIPP qu'ont été jadis donné aux régions pour les infrastructures et qui ont été acceptées par la Commission européenne dans le cadre effectivement d'un travail qui a essayé de le précédent, et encore, le précédent gouvernement, l'avis est défavorable mais il est ouvert à la suite du travail que feront les territoires avec le ministre d'État, l'écologie, et son secrétaire d'État, donc je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, dans d'autres textes que ceux de projet loi de finance de cette année. Merci monsieur le ministre des explications de vote Monsieur rénale. Oui, Monsieur le président, Monsieur le ministre, oui, je crois, nous avons tous entendu cet argumentaire qui est tout à fait, tout à fait pertinent de d'avoir une réflexion sur exactement ce qu'il faut. C'est à moi, ce que je crois c'est que on est, comme toujours dans une navette parlementaire ici et me paraît très utile, important de donner le signal, on peut certes se référer à vos propos, on peut aussi en votant un amendement finalement le marquer à cette étape de bras de la navette parlementaire, bon il n'y aura pas au-delà si entre temps il y a pas une solution qui a été négocié, nous le savons tous savaient, le gouvernement, mais moi je vous propose, à ce moment-là, une proposition à l'ensemble de de mes collègues qu'on ne se rassemble sur un seul amendement et je vous proposerai celui de notre collègue l'avare de Serrault qui me paraît le plus le

Merci, cher collègue Madame Goulet pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président du ministre Jacques là moi j'ai bien, j'ai bien compris les observations qui avait été faite en ce qui concerne la faisabilité des dispositions qui sont proposées, mais en même temps tous ces schémas sont relativement récent. Ils émanent en partie de la loi notre et donc à la fois leur mise en place et pas forcément bouclée et et en même temps les besoins qui suscite pas forcément non plus évalué, donc moi je je comprends un peu l'hésitation et je pense qu'il faut déjà laissé ces schémas se mettre en place, sachant le temps que ça prend déjà aux acteurs de terrain, de mettre en place des successions schéma on va déjà commencer par les et puis on verra ensuite, me semble-t-il la fiscalité qu'il faut il y appliquer néanmoins les amendements qui ont été déposées, l'ont été sur tous les bancs, donc doivent probablement venir d'une aspiration commune mais, mais moi je suis très prudente en ce qui concerne les schémas parce que dans ce pays, on a tendance à faire des schémas et des structures plutôt que de régler les problèmes, donc je maintiendrai sur ces amendements. Merci monsieur Huchon pour explication de vote. Oui, Monsieur le président, Monsieur le Ministre, vous savez très bien été rappelé tout à l'heure l'an passé, ici même, nous avons débattu du même sujet avec une quasi-unanimité, sénatoriales. Donc, un gouvernement et à l'époque, les objectifs étaient les mêmes rénovation par exemple d'environ 500000 logements par an. Et puis ça l'objectif n'a pas été atteint mais c'est logique, il ne suffit pas de décréter et puis de ne pas mettre ensemble les moyens, vous avez là un amendement qui est, je dirais non seulement une répétition d'une amélioration de la démarche qui a été faite l'an passé, vous avez une ambition qui était affichée par le gouvernement, qui d'ailleurs hier, ce qu'on avait pas au début de la discussion du projet de loi de finance le ministre à la fois de la cohésion des territoires et de la transition écologique et solidaire, a souhaité préciser les ambitions, hé bien, comme l'a dit Claude rénal et comme on le dit tous, c'est le moment de 6 mètres de faire est de travailler ensemble et de mettre Les moyens si vous ne mettez pas les moyens. Vous allez avoir, vous allez être pris en effet de ciseau avec cette fameuse hausse très importante de la fiscalité qui sera donc vécu que vous le vouliez ou non, comme une punition, et donc en mettant les collectivités soulever la double autorité finalement des régions avec le sera d'être le schéma régional de cohérence climat-énergie et puis les a intercommunalités qui sont, eux, à la tête également, qui ont la possibilité de de mettre en oeuvre ces démarches au service, à la fois du climat et de l'énergie, hé bien à ce moment-là, le gouvernement aura accompagné la demande de signal qui répond en même temps à la constitution faisons vivre faisons vivre cette république décentralisée, sinon ça veut simplement dire que la fiscalité auto service uniquement de l'État qui ne donne pas les moyens aux collectivités territoriales, quand bien même elle vous demande à la quasi-unanimité de travailler ensemble, hé bien Monsieur le ministre ici ce matin, je pense qu'on va vous dire chiche, on y va et fait avec nous.

les propos de de de notre collègue sont qui vient de s'exprimer, mais on est en ajoutant quelque chose en réponse à une intervention précédente les plans climat-énergie territoires sont apparus dans la loi, si je ne m'abuse, d'abord en 2004, rendu obligatoire en 2012 pour un certain nombre de collectivités et on a vu que parce que c'était pas financer un bon nombre de collectivités collectivités en avait adopté mais ne l'avait pas mis en ne les avaient pas forcément mises en oeuvre que d'autres ne l'ont même pas adopter, donc on a besoin effectivement d'un accompagnement réel parce que sinon les nouvelles collectivités qui sont maintenant obligés, à leur tour, de les mettre en avant, se met dans les pas de de celles précédemment, donc on a effectivement besoin

Oui, merci Monsieur le Président, le seul ministre, chers collègues, concernant, je dirais les différents amendements qui ont été déposés, je rentre je me rallye-raid naturellement à l'avis de la Commission et l'amendement aussi de notre collègue Madame Lavarde c'est réellement c'est vraiment des problèmes de société parce que ça fait très longtemps qu'on parle du développement durable et nos collègues qui font partie de la commission développement durable ça beaucoup mieux que moi et ont aussi beaucoup travaillé en liaison avec aussi les les autres commissions, mais je crois que ces débris D D des des problèmes de société alors sur les chemins, le plan climat la loi de transition énergétique et des textes qui existe depuis de nombreuses années, qui certes évolue avec de nouvelles dispositions, mais sur le terrain, je dirais dans le nous département respectif, on voit le la, un petit peu, on est toujours dans ce problème d'empilement de structures qui décide qui paye naturellement et se pose quand même vraiment des problèmes de complexité et et chemins, je dirais, dans lequel il y a une relative concertation, il faut aussi du temps de la compétence, mais aussi avoir une une vision globale, d'ensemble parce que il s'agit, pas que les chemins soit réalisé et après malheureusement reste lettre morte, comme on dit, et c'est malheureusement souvent le cas de de les filer l'efficacité, l'efficacité et les réalisations concrètes parce que Moralité, on attend du concret on, on, on sait qu'il faut faire des économies partout que le développement durable est une priorité, les énergies aussi réellement des des gros problèmes, on les voit avec les difficultés des chemins aux Liens aussi il y a les pour, il y a les contres c'est c'est vraiment des sujets de société et et après en terme de fiscalité et de moyens financiers, voilà, mais je me rallieraient à ceux à l'amendement de notre collègue jour merci. Merci Madame Lavarde pour explications de vote. Juste pour dire à monsieur le ministre, que par le vote de cet amendement, il donne les moyens de d'avoir des illustrations concrètes auprès des citoyens de l'augmentation de la fiscalité sur la TGAP et de ne pas en faire une fiscalité punitive mais une fiscalité qui va au service de la rénovation des bâtiments et je parle aussi à l'ancien maire, vous savez combien il est onéreux de remettre aux normes énergétiques et d'éviter d'avoir des passoires, les les petits oiseaux quand on a par exemple des mairies qui sont situés dans des bâtiments classés.

Merci Monsieur Ruquier monsieur. Oui, 3 observations : la première observation, j'ai bien entendu les remarques du rapporteur général et du ministre sur le fait que tout cela a un coût, mais la vérité c'est que le coût, il existe déjà, c'est pas la question, la question c'est qui supporte le coût qui existent déjà aujourd'hui, c'est ce sont les EPCI et les régions, ce qu'on propose, c'est que l'état y participent, voilà, ça c'était ma première observation, la 2ème, je pense, bien entendu, de la bonne volonté du du gouvernement, je pense que c'est amendement peut l'aider

à mon amendement, mais j'ai lu l'amendement Madame qui me semblent effectivement comme l'a dit un tout petit peu plus complet puisqu'il précise pour la métropole lyonnaise note et et la et et Paris donc je retire effectivement mon abonnement au profit de celui de Madame.

Qui est contre qui s'abstient. Donc il est il est adopté, donc il fait tomber tous les autres amendements en discussion commune.

positive, donc, cet amendement vise à attribuer aux collectivités locales une partie des moyens budgétaires récupérés par l'État via la hausse de la fiscalité écologique, donc c'est exactement la même philosophie mais pour accompagner les territoires à énergie positive

de la commission pardon. Même chose, bon c'est sur des appels à projets même problème de répartition que constater précédemment, donc même avis malheureusement défavorable. Monsieur le Ministre défavorable. Donc il y a pas d'explication de vote donc sur l'amendement 457 avec un avis défavorable de la commission de l'avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté l'amendement 186 rectifier bis Madame Boulet. Oui, Monsieur le Président, c'est un amendement Monsieur le Ministre, auquel tient beaucoup Françoise Ferrat il s'agit de répondre à l'objectif de moins 2 degrés de d'augmentation de la température de la planète, il convient de promouvoir des énergies renouvelables et de décarboner l'énergie cet abonnement contribuer à cet objectif environnemental en veillant à aider les entreprises pour le remplacement de leurs véhicules fonctionnant aux énergies fossiles, le parc des flottes d'entreprises fonctionnent au diésel, environ 90 pourcent par des véhicules fonctionnant avec des énergies renouvelables pour cela, il est proposé d'octroyer l'exonération de taxe sur les véhicules de société pendant une période de 12 trimestres aux véhicules fonctionnant au super éthanol E85, il s'agit d'appliquer à ce biocarburant un régime qui existe déjà pour les véhicules fonctionnant gaz naturel carburant ou au gaz de pétrole liquéfié, c'est l'objectif de l'amendement présenté par Madame Ferrat. Merci, monsieur le rapporteur général. Exonérés de taxes sur les véhicules société ça a un coût, on peut comprendre l'intérêt en effet de d'inciter les flottes d'entreprises à passer à des carburants. Meilleur pour l'environnement et donc notamment avec du super-éthanol 10 85, bon, il faut simplement le principal coût pour une entreprise, c'est sans doute le coût d'utilisation parce que les flottes d'entreprises roule beaucoup

contre 66,29 euros par litre pour l'essence donc le différentiel est assez significatif, les entreprises ont tout intérêt à utiliser ce type de véhicule car elle s'y retrouvent dans le coût à la pompe en fait d'un coût d'utilisation, donc c'est ça ne paraît pas nécessaire que la perte de recettes : avis défavorable. Monsieur le Ministre. Monsieur le président, la sénatrice, la difficulté, indépendamment du fait que ces véhicules ont déjà une une fiscalité qui qui leur est propre, est plutôt favorable, les véhicules que vous évoquez peuvent rouler indifféremment avec le le carburant que vous citez, mais aussi avec les sens sens et nous sommes pas convaincu puisque votre sujet effectivement nous partageons, c'est-à-dire à la protection de la planète et la lutte contre le changement climatique, cette mise en place de vie, ce qui a été, vous nous proposez atteignent l'objectif que vous évoquez, puisqu'on peut y mettre aussi, de l'essence et puis le 2ème point rapidement, c'est que le PLFSS 2018 en matière de de TVS pourra véhicules mis en circulation à compter de 2015, 2011 dans la législation actuelle,

Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, les collectivités, départements d'outre-mer font face à des enjeux majeurs pour la cour, la continuité et le développement du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, tant sur le plan financier que sur le plan technique et environnementale aussi ce contexte conduit à ce que l'augmentation de la TGAP ne soit pas incitative mais pénalise les Budgets des collectivités malgré les stratégies menées dans ce domaine

et ce n'est pas le cas dans le c'est territoires ultramarins sachez par exemple qu'à la Réunion 75 pourcent des déchets produits par les ménages sont enfouis en l'absence de mode de traitement et du fait de l'éloignement géographique ainsi la TGAP réduit la capacité d'investissement et accès à la accentuent leur temps déjà pris la modulation, demandez donc l'harmonisation avec les taux pratiqués en Guyane et à Mayotte, le temps de rattraper le retard dans la mise en oeuvre des outils multi-filières sur le territoire de la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, telle est le monsieur le ministre, le sens de cet amendement. Merci, monsieur le rapporteur général avec la commission.

Merci Monsieur président laisser entrer ses installations de stockage de déchets non dangereux situé à Mayotte éoliennes nécessite des tarifs réduits. De la TGAP plus importants que ceux dont bénéficient ces mêmes installations, ce qui en Martinique, Guadeloupe et la Réunion et vous posez donc d'harmoniser les tarifs entre ces ces territoires, des installations de stockage des déchets non dangereux à Mayotte et en Guyane sont sont plus importants que ceux dont bénéficient ces mêmes installations situées en Martinique, Guadeloupe et à la Réunion, je me permet d'être en photo dans votre présentation factuelle et une telle harmonisation que vous proposez réduirait donc le caractère incitatif de la TGAP déchets dans ces territoires qui ne serait donc pas cohérent avec les orientations de la politique gouvernementale, on propose un retrait que vous puissiez continuer à travailler cette question si vous souhaitez avec Madame Girardin, dans le cas des assises Outre-Mer avec le volet écologie et transition énergétique si vous souhaitez sinon un avis malheureusement défavorable. Monsieur ma grand-. Explications de vote. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre Monsieur rapporteur général la collègues j'ai cosigné cet amendement avec ma collègue, bien que sachant que il ne concerne absolument pas la collectivité que je représente, mais je suis aussi présidente délégation et la problématique des déchets en outre-mer et d'une problématique de fond qui ne peut pas trouver les solutions aussi facilement qu'elle le trouve en métropole, le sujet est tellement important que mes collègues ont unanimement souhaité qu'un débat de fond soit menée sur la question, malheureusement, les urgences de notre programme, nous oblige à reporter les résultats seront connus pour 2019 2019 nous sommes d'engager les résultats sont connus pour 2009 ce que demande ma collègue en fait. Eh bien réel stade il y a une pénalisation de la d'une d'une situation qui est déjà en situation défavorable, donc moi à titre personnel, ce que je vous dis, j'ai bien entendu la demande de retrait néanmoins si ma collègue maintenait son amendement, je pense que je l'ai cosigné je le voterais et non seulement je le voterai mais j'aimerais vous inviter à en faire autant, parce que je, j'estime qu'elle ne demande qu'un sursis de d'autant qu'il y a un engagement de ces collectivités à trouver une solution pérenne et durable.

La Martinique ont certes bénéficié d'une baisse avec la mise en place d'un coefficient multiplicateur de 0 75, mais cet effort rétrécissent visant pour mer permettent la réalisation des équipements indispensables pour sortir du tout en enfouissement en fait, vous savez que nous connaissons les prix élevés des matériaux implanté qui multiplie le coût des projets et pour faire face à à la création de nouveaux équipements,

je l'entends tout à fait la seule difficulté, c'est que si vous veniez à adopter cet amendement, il y aurait des territoires qui gagnerait territoire qui perdrait, puisqu'il aurait moins d'effets incitatifs pour d'autres, puisque vous proposer une harmonisation donc, malheureusement, je ne crois pas que l'adoption de cet amendement réglerait un problème dont je ne n'ignore pas au gouvernement, n'ignore pas l'intérêt,

ce qui pratiquent avant ces sujets de transition écologique et de déchets auprès des collectivités ultramarines, il me semble aussi qu'une réunion spécifique serait intéressante, je ne suis pas sûr que la votre option de cet amendement même qui soulève un problème et j'entends le dialogue que vous souhaitez réglerait le problème au contraire il accentuerait pour d'autres collectivités que celle que vous défendez manifestement. Monsieur le Ministre, donc je vais mettre aux voix l'amendement 267 pour lesquelles la Commission demander l'avis du gouvernement, qui a demandé le retrait qui sinon était défavorable, donc on a des avis défavorables qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Donc il est adopté, je mais au voit l'article 9 terre. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient,

Oui, merci Monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, c'est un amendement qui précise que le carburant biodiesel au bioéthanol des 10 a été introduite dans la nomenclature des carburants Soumiya à la à la TGAP depuis cette année, hein, c'est la première fois en 2017 effectivement, et donc il est proposé par cohérence de pouvoir introduire cet amendement aussi un des chefs du du du code des douanes, de façon à ce qu'il soit aussi redevables de la taxe supplémentaire à la TGV TGAP, de façon à inciter à ce que la filière agro-industrielle française puisse se développer, effectivement, je crois que nous avons dans notre pays, des agriculteurs qui sont en capacité de pouvoir apporter des compléments à nos carburants, voire même pour le bicentenaire de pouvoir apporter totalement la la ressource pour pour le carburant, donc, il convient d'encourager ces filières, de façon à réduire notre dépendance énergétique vis-à-vis de l'étranger.

Monsieur le président, il vient d'être défendu mais j'insiste : Paris primitivement sur le fait qu'il faut conforter cette filière, ça fait partie d'un subtil quilibre Inde de l'engagement d'une profession de d'une vision très, je dirai très positive et très pertinente vis-à-vis de l'environnement et si je puis dire, quitte à l'émergence, ainsi, je l'ai dit encore cette nuit, hé bien de tout ce qui présidera ce qu'on appelle la chimie verte.

D'après les a. Formation et l'analyse qu'on a pu en avoir l'article 9 quater telle qu'il était adopté par les seuls nationale mais si on ne tourne pas en l'état, donc je c'est la raison pour laquelle le garnement a déposé semble-t-il ce matin à un amendement qu'on n'a pas eu le temps de l'examiner en commission qui nous être présenté dans un instant et qui nous semble à l'heure qui nous semble à l'heure actuelle à régler les problèmes rédactionnels et moins d'applications que pose la la rédaction actuelle, l'article 9 quater si c'est le cas, j'éviterai les auteurs de ces 4 amendements à se rallier à l'amendement du gouvernement

Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. ce qui a évoqué les sénateurs, donc je serais assez d'avis Monsieur le Président, que votre assemblée adopte 613 en répondant favorablement à la demande de monsieur le rapporteur général. défavorable sur les autres puisque le rédactionnel 613 et est conforme, me semble-t-il, à la ce souhait de l'Assemblée et sécurisant juridiquement. Merci, Monsieur Bizet pour explication de vote. vote. Monsieur le président Monsieur mis mes chers collègues, je, je suis absolument désolé, cet amendement, qui se veut rédactionnel ne me plaît pas, pour la bonne unique raison, c'est que il souligné véritablement de la définition que souhaite donner le le code des douanes, le code des douanes et très explicite les TGAP ne peut être que sur des produits précisément identifiés par référence à leur indice dans le tableau B du I de l'article 265 du code du code des douanes, or l'amendement rédactionnel du gouvernement est beaucoup trop tôt ouvert, je ne voudrais pas imaginer qu'au travers de cette ouverture, on nous amène tout doucement de Manhattan et bien des carburants issus de la filière huile de palme, ce serait tout je dirais sauf désagréable vis-à-vis de l'environnement tout sauf désagréable vis-à-vis de de de la filière, je dirais, gros agrobusiness du du nord de la France et je ne vois pas pourquoi au travers de cet amendement rédactionnel on on rentre dans une définition beaucoup moins précise que l'exige le code des douanes. Chers collègues, monsieur le rapporteur général. C'est un peu technique, c'est vrai, c'est pas forcément très compréhensible, comme on vient je viens découvrir l'amendement 613 ans n'a pas du tout le temps d'examiner en commission et ni même de l'expertiser et donc la seule

Monsieur Ligier, vous êtes déjà intervenu en explications de vote, donc je ne redonne pas la parole, explications de vote donc. Après est-ce qu'il y a d'autres explications de vote. Donc sur ces amendements. Compte tenu de l'amendement du gouvernement 613 pardon, monsieur le ministre vous apporter, mais c'est juste. Pour répondre à l'interrogation de Monsieur sénateur Bizet, enfin il y a déjà un décret qui existent, ce qui relève des biocarburants et ce qui n'est pas 16 pas corrigée par l'amendement rédactionnelle du gouvernement, donc il y a pas de changement de philosophie, donc, ne vous en inquiétez pas et je précise le rapporteur général, une nouvelle fois le et 10 hé bien concerné.

la rédaction du gouvernement et et plus cohérente et plus favorable à l'ensemble des arguments évoqués. Monsieur qui a pu explications oui je compte tenu de 2 explications de du ministre et je prends acte de ces explications, je me rallie à son amendement, je retire le bien du coup.

pour la Commission. Pour la Commission, servi de sagesse. Allez, allez, de sagesse de la Commission. Donc, le 147 478 et 531 jamais au bois qui est pour.

simplement simplement d'exclure le des 95 de l'assiette de la TGAP car tout simplement il ne contient pas de carburant fossiles, faut-il rappeler ici, Monsieur le ministre et vous avez, vous l'avez évoqué très largement hier soir que on pouvait agir par la TGAP, or l'objectif de la TGAP, taxe générale généralisée sur les activités polluantes, c'est d'inciter à l'incorporation de biocarburants vertueuses du point de vue écologique agricole, alimentaire et satisfaire l'économie locale voilà Musso me là sur un sujet de innovant qu'il faut promouvoir. Merci, cher collègue, le 149 rectifier Monsieur

écoutez, signé par amitié, défendu par avance par les collègues qui l'ont déjà défendu puisque c'est le même sur les sur tous les bancs, c'est un amendement auquel tenez madame ferraille qui a déjà été défendue par plusieurs collègues. Merci pour votre amitié. Monsieur Lalonde. Le 342 rectifier. Défendu aussi Monsieur Capulet 368 rectifier. Il est défendu, je vous précise juste que c'est un carburant qui est utilisé dans plusieurs villes de France et notamment à Angers, qui en tire toute satisfaction et qui émet beaucoup moins de particules et de gaz à effet de serre. Merci, monsieur le rapporteur général l'avis de la Commission sur ces 5 amendements.

merci. Défavorable du gouvernement. Donc on a une demande de retrait de la la Commission oui mais ce qui perce. Je je maintiens, je maintiens cet amendement parce que ne nous mettons pas dans une situation de fragiliser un développement qui sera porteur, demain, on peut pas supprimer le gasoil et en même temps ne pas donner de substitution, or le 95 est un élément qui ne comporte pas d'éléments fossiles et qui est vertueux, je suis désolé, je le maintiens.

Qui est contre. Qui s'abstient ils sont adoptés. Nous passons un amendement dont nous avons déjà parlé de 613 du gouvernement Monsieur le Ministre. Je crois qu'il a déjà été défendue. Déjà défendu monsieur le rapporteur général l'avis de la commission. Sagesse

Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté. Nous poursuivons avec 4 amendements identiques, le 148 rectifier monsieur Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, effectivement c'est un amendement qui concerne le sans carburant. Entièrement renouvelables qui constitue à notre sens, une véritable alternative au diésel classique et qui permettra d'atteindre les objectifs ambitieux que la France doit se doter pour réduire sa dépendance aux carburants extérieur et donc il s'il s'agit de permettre obéissante d'être inclus dans le de 2 permet de l'émission de certificats pour le PS, sans, sans pour autant que ce carburant n'est à subir le la la taxe additionnelle sur les activités polluantes puisque il s'agit pour nous d'encourager totalement l'activité agro-industriel en France, comme l'a évoqué fort justement Jean Bizet tout à l'heure, c'est un enjeu que l'on considère comme majeure et donc il est nécessaire que l'on mette en place des outils permettant à ces filières de véritablement émergé d'être compétitive aussi par rapport au au carburant plus classique, sinon nous ne nous ne répond pas à développer de véritables filières industrielles en ce sens dans notre pays, ce qui est pourtant nécessaire pour développer l'économie ensuite assurer des ressources pérennes pour

organisée ce que elle ce qu'elle souhaite et loin de là, l'idée du Grand Nancy intéressé mais l'amendement du gouvernement satisfait ce qui vient dire, Monsieur le Sénateur, est satisfait, même si les rédactions ne sont pas identiques beaucoup d'amendements, 2 de vos collègues parlementaires, donc il ne m'aurait semblé assez logique qu'une partie d'entre-temps avec l'amendement du gouvernement mais sinon je pense qu'on en discutera en vous disant que c'est déjà satisfait partisan, parce que vous avez adopté. Commission par rapport aux amendements suivants.-ce que l'amendement 613 du gouvernement qui a été adopté ce qu'il fait et Alors 2 minutes de suspension de séance.

Chers collègues, la séance et reprise donc nous poursuivons la discussion commune.

Il a été défendue, c'est, c'est exactement le même rendement de manque, celui qui a été présenté, c'est sur le blessant. Merci, Monsieur Bizet pour le 479. il a été défendu mais je précise en plus si vous voulez que cet amendement permet d'être en cohérence avec la directive 2009 28 qui permettrait plus aisément à la France d'intégrer les objectifs européens de 10 pourcent d'incorporation d'énergies renouvelables dans le secteur des transports à horizon 2020.

Merci donc l'avis de la Commission, monsieur rapporteur. Je précise bien pour la bonne compréhension de l'Assemblée, c'était un peu compliqué que le 9 quater telle qu'il a été votée à l'Assemblée ne tournait pas, ne fonctionnait pas, donc c'est la raison pour laquelle le garnement à déposer un amendement, je regrette simplement qu'il arrive à la dernière minute, ce qui ne pas le temps, l'expertise et on n'a pas pu vérifier, sur le fond, la compatibilité avec l'amendement qui a été adopté et proposée par Jean Bizet, donc sans doute légitimement formellement les 2 rédactions ne sont pas compatibles,

porte le nom baissant mais contenu du du de date Corporation dans la filière diésel qui est fixée à 7,7 pourcent ça aboutirait non seulement exonérés de TGAP mais ça irait au-delà et ça créerait des avoirs fiscaux de TGAP donc déserts fiscaux que ensuite évidemment, il peut être commercialisé donc épaulé par les distributeurs, donc c'est pour ça qu'on était plutôt défavorable sur ces amendements qui vont au-delà d'une simple exonération. Merci monsieur le ministre pour la vie du mur gouvernement défavorable. Oui, le président Guillaume pour explication de vote. Le président, monsieur le ministre, les amendements de Jean Bizet du gouvernement sont ni parallèles ni antinomique. Ils ouvrent d'autres portes différemment, je pense que ces amendements juridiquement pour notre assemblée ne tombe pas, moi, je me sens mais, chers collègues, qu'il faut les voter, et dans la navette, on verra comment tout cela pour pouvoir entrer parce que ce que je ne voudrais pas non mais, chers collègues, ce que je ne voudrais pas c'est que, en décidant qu'il tombe et qu'ils ne sont plus là, vu qu'il a manqué de l'expertise de un moment d'expertise pour l'amendement du gouvernement on soit privé dans certains thèmes, donc on est en première lecture, je pense que c'est pas très grave, me semble-t-il, et dans la navette, Jean Bizet, qui est un expert avec les administrateurs de la Commission, le président du gouvernement verront ce qu'il va mieux dans une peut-être nouvelle rédaction

Merci madame Prima pour explication de vote. s'perd un peu entre la TGAP sur le B 10 le baissant le B chez pas quoi le bioéthanol le niveau d'incorporation, on est complètement perdue, moi je, j'ose le dire, en ayant pourtant un petit peu regardé le le sujet donc j'appelle de mes voeux des clarifications, ce qui est polluant, hé bien il y a la TGAP, ce qui est pas polluant et qui, énergies renouvelables, issus de l'agriculture etc, n'est pas taxé et puis voilà, enfin, je pense qu'il faut revenir sur des choses qui sont des choses assez simples, donc peut-être faut-il y a effectivement voté ces amendements pour ouvrir la discussion et assure que cette discussion soient faites, je sais pas si le PLR c'est le meilleur moment, mais en tout cas un peu de clarification de vos voudrait bien. Merci monsieur Karoutchi pour explication de vote.

je je m'adresse à Alain Richard, comme à tous ceux qui vont travailler sur la réforme constitutionnelle est-ce que c'est du niveau législatif est-ce que c'est du niveau du Parlement la de voter sur est-ce que le B 17 heures entrée ou pas, franchement c'est. Totalement en dehors du domaine législatif, mais comme on s'habitue à se dire tous ensemble que de toute manière plus vaut mieux que moi, on continue de voter des amendements que l'année suivante on contredit d'ailleurs avec la même détermination, ils ne sont pas plus du domaine législatif, l'année suivante et on continue, et là, franchement, alors on en est à dire maintenant, il y a un amendement du gouvernement qui vient d'être votée, mais alors comment au millimètre auprès, il est pas exactement sur les amendements qui eux-mêmes ne sont pas législatif mais sont du domaine réglementaire, mais ça fait rien, c'est pas exactement les mêmes, et j'entends président Guillaume qui dit pas très grave, première lecture on peut vous avez raison mais franchement on se dit nous-mêmes, entre nous, nous ne sommes pas dans le domaine du législatif, nous entrons dans un débat d'une technicité tels que, par définition, pardon, mais l'essentiel des parlementaires votent comme leur groupe, tout comme le rapporteur, sans trop savoir mais si

si on pouvait messieurs, président de la commission des finances, le rapporteur général et après nous, faire en sorte que les amendements qui ne sont pas du domaine législatif n'arrive pas au Sénat. Merci, mes chers collègues monsieur Longuet pour explication de vote. monsieur le président Monsieur Luis, mes chers collèges, je voterai ces amendements pour les raisons excellente que Didier Guillaume, a présenté, mais pour répondre à mon excellent collègue lui aussi Roger Karoutchi il est vrai que nous donnons le sentiment de faire du travail de commissions en séance publique, ce qui est relativement coûteux parce que la séance coûte plus cher que la commission, cela étant, le débat est utile et s'il ne vient pas en séance publique, je constate qu'il n'a pas eu en effet dans cette affaire de carburant, il faut distinguer 3 problèmes qui n'ont rien à voir. Avant d'être un carburant le diésel est un moteur inventé par Rudolf Diesel et ce moteur a des singularités qui lui permettent de tirer un meilleur parti du carburant carburant que ce carburant soit ou qu'il soit végétal, la France a fait le choix du diésel, non pas pour embêter les petits oiseaux, mais pour une époque nous étions, nous le sommes d'ailleurs toujours lourdement déficitaire sur la balance des combustibles, le diésel a l'Avantage de consommer moins pour des kilomètres parcourus et donc toute la politique fiscale en faveur du carburant du moteur diésel du moteur diésel procédait de l'idée qu'on consommait moins pour avoir un service supérieur. Est apparu à juste titre la préoccupation environnementale : on peut remplacer pour alimenter un moteur diésel dès le le l'origine fossile par l'origine végétale, c'est ce que propose l'ensemble des des amendements qui qui vont de de B 25 à abaissant j'en suis convaincu, là on est dans le domaine de la technique de la commission des finances, il est vrai que ce travail si nous avions eu l'amendement plutôt, nous aurions pu l'engager, secret, enfin 3ème problème, c'est que le végétal n'est pas ne signifie pas pour chacun d'entre nous, exactement la même chose, le végétal lorsqu'il procède de l'huile de palme soulève à juste titre des préoccupations légitimes sur le plan, hein, de la balance des paiements et surtout de l'environnement car les végétaux du du traité européen son sont produit dans des conditions qui sont connues et acceptées les végétaux, lui, l'issue de la palme est produite dans des conditions que je qualifierais pour le moins d'incertaines et c'est exactement ce débat que nous avons sur ces 3 points, sauvons le moteur diésel du carburant qui respecte l'environnement, choisissons le là où on sait comment il est produit, c'est la raison pour laquelle je soutiens ces amendements. Et merci, cher collègue, Monsieur Bizet pour explication de vote. monsieur le président Monsieur mise, mes chers collègues, je pense malgré tout que ce débat dont on n'avait pas imaginé, je dirais, la dimension et l'issue nous permet d'élever quand même le débat sur un sujet, c'est vrai, un peu complexe, un peu technique, qui est celui de des biocarburants, donc moi je souscris à la proposition de Sophie Primas et Didier Guillaume, de remettre un petit peu tout à plat et c'est l'occasion où je pense, plus rationnel, plus rationnel, peut-être que ce soit en commission mais nous y sommes là mais je crois qu'il faut avoir en filigrane 3 ou 4 idées claires au-delà de ce qu'a dit fort je dirais fort justement notre collègue Gérard Longuet que nous sommes là en face de carburant renouvelable que c'est dans l'air, non seulement du temps et si je puis dire, dans le droit fil des recommandations de la directive 2002 2009 28 que nous sommes là, également, à la veille d'une lisibilité accrue d'une filière naissante qui est né il y a une dizaine d'années, la filière je dirais oléoprotéagineux The et qui a demandé plus d'un milliard d'euros d'investissement pour la profession agricole qui a 3 facettes : on l'a dit depuis cette nuit encore, ce matin, 3 facettes assez extraordinaire, hein, de produire du carburant de produire des protéines végétales garantir une équilibre de notre balance commerciale et 3, on ne le sait pas encore suffisamment ça produit également ce qu'on appelle du glycérol, c'est-à-dire que nous sommes à la veille d'ouvrir toutes important en matière de d'énergie donc moi je suis ravi que, à l'occasion de ce débat, on puisse mettre à plat tous ces biocarburants l'amendement 478 que j'avais proposé, si vous voulez, était beaucoup plus précis et répondait à une question essentielle qui, c'est-à-dire le le le code des douanes l'amendement du gouvernement 613 laisser la porte entrouverte de nous a dit que non, à la production, avant tout, il y a l'incorporation d'huile de palme alors il a dit que c'était pas spécialement explicite mais si vous voulez, c'est quand même assez dangereux ont une grande confiance n'exclut pas une petite méfiance donc moi je continuerai à imaginer de voter les différents amendements mais il faudra qu'on mette toute la filière biocarburants à plat. monsieur le président de la commission des finances. Oui, j'ai souhaité m'inscrire dans ce débat après l'intervention de notre collègue Karoutchi car s'il est évident que le débat dans lequel nous sommes est un débat d'une relative technicité, il n'en reste pas moins que la définition de la société du taux de l'impôt, c'est une prérogative du Parlement depuis l'ancien régime, donc je pense que nous avons quand même là un sujet dont on voit bien gérer l'importance je dirais d'effets économiques sur notre monde agricole en particulier, donc on ne peut pas s'en dessaisir j'irai dans son principe et donc il faudra bien qu'on rende dans cette technicité, la difficulté devant laquelle nous sommes, c'est que est survenue assez tardivement hier après-midi, autant que je le sache, un amendement du gouvernement qui modifié assez substantiellement l'ensemble du dispositif et que nous avons pas eu le temps d'y travailler réellement de façon approfondie, donc ça renvoie plutôt au débat qui s'ouvre après les déclarations de monsieur le ministre sur la question de la procédure vrai parlementaire sur la loi de finances, donc voilà, on va reprendre ce travail mais effectivement la solution qu'a évoqué notre collègue Guillaume qui consiste finalement à adopter un certain nombre de dispositifs au travers des différents amendements qui n'ont pas été déclarés en discussion commune et qui donc ne se tiennent pas les uns les autres, on va aller voter s'il y a un espace de contradiction ou s'il y a, je dirais, des trous dans la voilure, hé bien le processus le processus d'élaboration de la loi avec une seconde lecture la navette la CMP etc régule rend cette affaire on va veiller les uns et les autres, de façon à ce que la question respect pas en l'état où nous allons le laisser dans quelques minutes, voilà ce que je propose. Si Monsieur le ministre.

huile de palme étaient concernés aujourd'hui avant même notre débat parlementaire dans le décret, j'ai évoqué tout à l'heure après il y a un autre débat il y a peut-être vers d'autres amendements qui évoque de retirer les carburants qui sont la base de, de, de, de, mais c'est pas le sujet de discussion de maintenant donc l'amendement du gouvernement ne permet pas un nouveau droit de faire entrer l'huile de palme dans ces carburants puisqu'ils y sont déjà, que ce soit bien clair entre nous et pour qu'il n'y a pas confiance et et de contrôle, qu'il n'y a pas de de de mésentente sur ce qu'on se souvient de d'évoquer entre. Monsieur Calvet pour explication de vote. Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, bon, ce débat est extrêmement intéressant parce qu'il permet, dans le cadre du budget d'affirmer un certain nombre d'orientations que nous voulons mettre en oeuvre et qui se trouve dans d'autres textes comme cela été évoqué tout à l'heure des objectifs de développement des énergies renouvelables et de véritable transition énergétique, il importe qu'effectivement nous puissions les traduire très concrètement dans dans les Budgets, ça amendement ne vise pas exonérés de TGAP, il vise à exonérer exactement de du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes pour éviter que ces carburants ne soient véritablement grevée d'une fiscalité pénalisante, donc c'est bien l'objet de de ces amendements, nous devons je crois très clairement affirmer que nous, nous voulons que dans notre pays se développe une filière de production des carburants, nous avons un commerce extérieur qui est particulièrement déficitaire à 34 milliards de déficit commercial au 1er semestre 2017 et nous n'arrivons à le résorber que si nous prenons les mesures qui permettent de développer un certain nombre de filières, nous avons par ailleurs dès les activités agricoles qui sont en grande difficulté pour un certain nombre dans notre pays, d'autres vont très bien, mais certains secteurs sont en difficulté donc il importe que nous puissions aussi permettre à nos actifs agricoles de pouvoir prospérer, c'est-à-dire de pouvoir mettre en place des productions qui répondent à de véritables enjeux et si demain la France peut non seulement réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur, mais en plus être exportateur de carburant et ainsi répondre aux objectifs de développement des carburants renouvelables et propres en Europe et dans le monde et donc mettre en oeuvre réellement les objectifs de la COP 21, hé bien je crois que nous aurons véritablement mener notre fonction de parlementaire en tout cas moi j'invite à ce que, à soutenir ces amendements.

monsieur le président, Monsieur le Ministre, on a pu constater en 2007, un détournement de la TGAP avec justement les importations de d'huile de palme donc ces huiles notamment n'ont pas de qualité vertueuse, puisqu'elle dégrade la qualité de l'essence sont incorporées aujourd'hui sans pouvoir améliorer la qualité des essences, elles sont là simplement par effet d'aubaine pour simplement profiter de la TGAP donc le l'objectif de cet amendement et de mettre fin à cette effet d'aubaine, tout simplement, en clarifiant que seuls les biocarburants explicitement mentionné notamment produit à partir de céréales françaises et d'autres plantes riches en amidon puissent justement prendre tout leur sens, voilà, c'était fait de Debanne doit être

et je remercie Roger Karoutchi au passage d'avoir d'avoir institué mon amitié et ma conviction endoctrine sénatoriales. Merci même voulait le 340 rectifier Bernard en. Monsieur le président, Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, l'objectif de la TGAP est donc d'inciter à l'incorporation de biocarburants dits vertueux d'un point de vue écologique agricole, alimentaire et doit favoriser l'économie locale. Or l'objectif que de cet amendement que nous présentons est de clarifier que les biocarburants sont les seuls pouvant entrer dans le Champ d'application de la TGAP, notamment les carburants, les biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon ou sucrière pour l'objectif de 7 pourcent dans les essence, que constate-t-on, on constate que 100 pourcent du HVO de type échéances sont essentiellement importés, ils sont utilisés en France et ils sont produits à partir de l'huile de palme, vous avez donc compris que cet amendement et donc de favoriser la production de biocarburants sur notre territoire, biocarburants qui seront de toute façon écologique et bien sûr agricole merci. Merci, cher collègue, monsieur le rapporteur. peut-être, donner un avis sur amendement j'juste expliquer pourquoi ce matin nous avons l'impression de faire un travail de commissions et et nous avons ces incertitudes, tout simplement parce que l'article que vous a mis dans l'article 9 quater déguisé si l'Assemblée nationale ne fonctionnait pas, ne tournait pas, pour être très clair, ça avait été signalée dès le 15 novembre dans le rapport de la commission, donc on l'avait dit, très concrètement, on est un petit peu de mal d'avoir pour avoir les informations nécessaires et procéder aux rectifications qui aurait permis que cet article 9 quater fonctionne pleinement et nous sommes aujourd'hui presque 9 jours après nous avons eu, il y a après midi tardivement l'amendement du gouvernement, donc c'est évidemment. Toujours la difficulté du travail parlementaire, je vous rappelle que le dépôt des amendements, c'était vendredi à 11 heures avec un examen en commission, à 9 heures une séance publique commence le lendemain et nous avons plus de 600 amendements, donc j'ai entendu ce qu'a dit Monsieur le Ministre, qui à nous appeler, et je le dis clairement comme l'a dit, l'instant, le président de la commission des finances, nous sommes prêts à travailler avec vous a trahi que nos homologues Monsieur Ministre de la commission des finances de l'Assemblée nationale pour regarder cette procédure budgétaire qui est folle, encadrée par des délais 40 jours à l'Assemblée 20 jours au Sénat et qui pose d'énormes difficultés pratiques pour travailler les un travail, il est l'être législatif sérieux et je ne parle même pas du PLFR que nous examinions des commissions qui sont encore plus désagréable des folles parce que nous sommes parfois, est amené à statuer en commission, alors même que nous n'avons pas par écrit le texte définitif de l'Assemblée nationale, c'est ce ceci ensuite les difficultés pratiques que nous connaissons les difficultés à porter un véritable jugement sur des articles parfois extrêmement technique, mais lourd de conséquences parce que nous sommes bien qu'on le veuille ou non, de la fiscalité, dont c'est le rôle 1er du Parlement de fixer les bases et les taux des impositions, donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle bon, on n'a pas, sans doute, ce matin, réalisé un travail absolument parfait, il faudrait revenir au cours de la navette alors sur les sur ces amendements depuis un petit peu différent, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas été mis en discussion commune puisqu'il s'agit, en clair d'exclure l'huile de palme. Du taux de prélèvements supplémentaires de TGAP applicable à l'essence et c'est vrai que la Cour des comptes dans son rapport annuel 2000 16 heures consacrées aux biocarburants a considéré que la montée en puissance des importations d'huile de palme qui sont évidemment en provenance d'autres pays que l'Europe du pays tropicaux a contribué à déséquilibrer les filières parce que c'est lui et souvent moins coûteuses que que les huiles comme l'huile de colza qui sont produits de de, notamment en France, donc c'est un vrai débat et il y a de fait une sorte de détournement de la TGAP dans la filière essence avec ces biocarburants

D'abord, Monsieur le Président, partager propos du président de la commission des finances et du rapporteur général sur la la révision finalement de nos études de texte financiers et épuisé les les arrivées tardives des amendements du gouvernement, j'imagine qu'effectivement ce n'est pas bien simple ni pour vous ni pour vos collaborateurs d'y travailler, soyez rassurés sur le fait que moi-même je les ai parfois très tardivement, ce qui est en rien une excuse, mais qui peut être une justification de devant vous, par ailleurs, sur l'amendement que que propose votre collègue, c'est un avis défavorable pour une mesure d'égalité, en effet, rien ne justifie que nous puissions de traitement pour des carburants qui respecte tous les critères pour lequel nous avons ici une discussion depuis tout à l'heure, devait-il des présentement, c'est-à-dire de ne pas encourager la corporation de carburant qui se produit dans des conditions nuisible pour environnement ce que vous évoquez, monsieur le sénateur est déjà satisfait, en effet, ne sont pas prêts au compte dans le calcul du tarif dégressif de la TGAP les cadrans qui ne satisfont pas aux critères à l'article L 661 5 du code de l'énergie, qu'ils soient ou non issus de l'huile de palme mais cette différence de traitement que vous souhaitez mettre mettre dans la loi, malheureusement, ne passerait pas le constat du Conseil constitutionnel ou les recours éventuels aucun avis défavorable. Donc jamais au bois le les amendements identiques 25 rectifier 184 rectifier bis et 340 rectifier qui ont reçu un avis de sagesse de la Commission, un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient ils sont adoptés. Nous poursuivons avec 4 mois en en en discussion commune le 23 rectifier monsieur Cuypers. Cuypers. Ce président, Monsieur le Ministre, oui, ça rejoint l'année les amendements précédente, contrairement à l'éthanol qui est défini dans la norme NEC 15 376 aucune norme aujourd'hui n'existe pour définir les huiles végétales Hydro-traité de type essence cela montre tout simplement que ce produit ne peut être contrôlé l'objectif de mon amendement et de mettre fin à cet effet d'aubaine que je rappelais tout à l'heure en clarifiant que les biocarburants produits à partir des 8 E acide, en particulier des usages acide de panne n'ont pas leur place dans l'objectif de 0 6 pourcent de biocarburants avancés dans l'essence, je rappelle que l'huile de palme, aujourd'hui c'est 1 des biocarburants incorporés, sur les 7 pourcent que produit la filière végétale française. Oui, Monsieur le président, Monsieur le Ministre, cet amendement auquel Madame Ferrat, tiens tiens beaucoup, c'est exactement celui qui a été défendue et en même temps on se retrouve encore sur cette sur cette même discussion avec les mêmes objectifs. Autour des des activités polluantes et aussi des un gros carburant vertueux, donc il y a rien à ajouter à ce qui a été dit, sinon à adopter cet excellent amendement. Merci Madame Goulet, le 341 rectifier monsieur Lalonde défendue. Le 551 monsieur pu. Oui, il est défendu, c'est la même, c'est le même objectif d'exclure les produits à partir du les acides de la fiscalité relative aux biocarburants. Merci, cher collègue, l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur. Tout à fait dans le droit fil des des précédents, cette fois-ci sur les acides, les huiles acides, la réponse sera un peu la même tout en entendant l'argument du ministre sur le problème d'égalité, donc il y a surtout d'un problème constitutionnel je, je, c'est la raison pour laquelle la Commission va pas être favorable, s'en remet à la sagesse du Sénat, eu égard aux risques évoqué le ministre. Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, l'avis du gouvernement défavorable, donc je 4 amendements 23 rectifier 183 rectifier 341 rectifier 551 avec un avis de sagesse de la commission à la vie défavorable gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient ils sont adoptés je mais au bois, l'article 9 quater, qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté. Après l'article 9 quater un article additionnel l'amendement 617 du gouvernement Monsieur, ministre. Oui, Monsieur le président, il s'agit en effet par cet amendement de maintenir le Champ d'application de la TGAP ses émissions polluantes et de conserver un niveau actuel des recettes pour cette composante de latex, en effet, le code des douanes prévoit actuellement que les installations de combustion soumise à autorisation dans la puissance thermique maximale est supérieur à 20 millions amateurs sont assujettis à la DGA plaider l'émission de substances polluantes dans l'atmosphère, en l'absence de la modification proposée, ce serait une perte de recettes monsieur de apporte général qui est évalué à 6 millions d'euros, qui serait constatés par l'État ainsi que par les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, dont une part importante des ressources vous savez provient d'abord libérateur de la TGAP, de surcroît, cette mesure assure le parallélisme des obligations déclaratives de ses installations avec celles soumises à la demande expresse du sénateur Karoutchi qui met en commander hier soir à l'État soit annuel des émissions et transferts de polluants, des déchets, c'est l'arrêté du 31 janvier 2008, mais vous savez, ça n'est pas le sinistre. Merci monsieur le ministre, l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur. Voici ce que pour l'assemblée qui s'est un moment nous est parvenue vendredi matin donc, malheureusement, après la réunion de la commission

Donc je m'en remets à la sagesse du Sénat ou alors provoqué option de séance mais je pense qu'on peut dans ce cas-là, ouvrent le dimanche, tout de suite un et si on examine chacun des si on fait une séance de la commission des finances sur chacun des amendements qu'ils étaient posées tardivement, je pense qu'on peut voir le dimanche donc, et même la nuit, tout ce qu'on veut, donc je m'messager du Sénat, vous êtes-vous. Merci, monsieur le rapporteur, donc sur l'avis sur l'amendement 617 du gouvernement avec un avis de sagesse de la commission qui est pour.

vous savez c'est un article qui prolonge le dispositif de suramortissement fiscal pour l'acquisition de véhicules de plus de 3 tonnes 5 qui fonctionnent au gaz naturel au bioéthanol est de 85 donc pour ces véhicules, ils ont un dispositif de suramortissement sur le fond, il apparaît pas particulièrement pertinent à la commission que le suramortissement soit utilisé comme le meilleur outil pour encourager les questions du véhicule, mais surtout nous n'avons, nous sommes dans la capacité totale de connaître le coût de cette niche fiscale et donc faute d'avoir pu obtenir, nous avions déjà posé des questions et dernière. Et. Le même traitement dont on ne sait pas si ça coûte, ça coûte, parce que c'est utilisé il y a pas d'estimation dans le bleu budgétaire donc, faute de pouvoir qu'avec le coût de la niche, hé bien on propose la suppression et Monsieur Bernard nous répond que c'est utile, il appartiendra de donner le chiffrage et dans ce cas-là, évidemment, je serai prêt à retirer l'amendement mais à l'absence de chiffrage, je propose de supprimer l'article 9 qui inquiète parce qu'il était prêt à la commission qu'il n'y avait pas d'utilisateurs de ces sur morte Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre pour l'avis du gouvernement simplement votre un moment un avis défavorable, j'espère que vous le comprendrez, puisque sur l'arrêt programmé Luis positive de ce soir dans 6 mois au 31 décembre 2017 que vous proposez, il y aurait une dynamique de développement qui serait freinée de cette. Hier, même si j'entends pour connaître la dynamique, encore faut-il connaître le nombre de personnes qui qui qui l'exploite, je l'entends bien volontiers, voilà donc un avis défavorable, peut-être monsieur le rapporteur général, puisque je n'ai pas les éléments de de ce chiffrage et j'en suis fort pourvu que l'on puisse en rediscuter en seconde lecture chiffrage à appui.

c'est que nous sommes à capable de savoir si il s'agit clairement d'une niche fiscale d'un Avantage fiscal qui est utilisé ou pas sur les dit ça concerne des milliers de véhicules, c'est utile, on est prêt à il faudra apprécier ça sur le fond

des réticences sans doute sur la pertinence des éditions Marty seulement mais à est-ce que le ministre nous apporter nous dire le nombre de véhicules concernés les les filières concernées : le nombre d'entreprises concernées, élus, ce qui va être d'apprécier la pertinence de dispositifs dans l'article, pour l'instant nous donne aucune indication. Et monsieur le rapporteur, monsieur le Ministre. J'entends tout à fait la la récrimination rapporteur général et je ne peux en tant qu'ancien parlementaire si permet de le dire, être d'accord avec lui donc ce que je vais faire, c'est que j'ai transformé mon avis défavorable en sagesse comme ça vous pourrez supprimé article gouvernement n'avait qu'à vous proposer effectivement des éléments vous allez demander légitimement demander institution et donc revenir en seconde lecture, peut-être avec des éléments que je n'ai pas non plus dans la possession donc à une sagesse qui irrespectueux, me semble-t-il, de vos demandes de.

Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur lui, chers collègues, voici donc un article qui nous propose de relever le plafond d'application du régime de la micro entreprise en procédant à son doublement, le tout pour un coût de 21 millions d'euros environ, on rappellera que le régime micro-entreprise peu concerner dans notre pays dès les 2 millions d'entreprises dépourvues de salariés que compte la France, dans cet ensemble, faut-il le souligner, nous avons notamment, et c'est là l'une des sources, des difficultés du RSI la longue cohorte des auto-entrepreneurs, plus d'un 1000000 100 1000 aujourd'hui, dont un bon tiers d'ailleurs n'a, n'a pas d'activité quant aux 2 tiers restants leur chiffre d'affaires est sans commune mesure avec le relèvement de plafond dont il est ici question. Parce qu'il faut tout de même atteindre 170000 euros de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas rien, ce qui fait que la mesure dont nous parlons avec cet article 10 devrait finalement privé l'État de 3 millions d'euros de recettes d'impôt sur le revenu, partagé entre environ 5900 entreprises soit un Avantage limité à 500 euros par an, la mesure pose certains problèmes de justice et d'équité, selon nous, on rappellera qu'avec un plafond de 170000 euros, certains entrepreneurs vont se retrouver avec un abattement d'office de 71 pourcent de leurs revenus, une absence de tenue de comptabilité et la poursuite de la pratique d'un prélèvement forfaitaire en matière sociale et fiscale avantageux ainsi à l'entrepreneur qui réaliserait 50000 euros de chiffre d'affaires n'aurait à payer que 145 euros d'impôt sur le revenu, la réforme n'est pas présentée comme la base d'un Avantage fiscal mais force est de constater que la situation des entrepreneurs individuels sera sans doute meilleure que celle des salariés, si elle est adoptée en l'état un salaire de 100000 euros brut par an, porte en effet aux alentours de 60000 euros de cotisations sociales et doit s'acquitter d'un impôt sur le revenu, autrement plus conséquents outre le donc la distorsion pouvant procéder de l'article 10 dans la situation des artisans, c'est aussi dans la comparaison entre actifs salariés et non salariés que la question se pose : nous pensons pour notre part que les entreprises n'ont pas grand-chose à gagner de mesures fiscales de ce type, la bonification des prêts accordés aux PME et aux artisans, les primes à l'installation semble, selon nous, des moyens aussi efficace de répondre à l'attente des artisans et commerçants individuelles, merci.

très critiques à l'égard de de l'article 10. Je ne paraît extrêmement sévère. L'article 10 non plus n'est pas une révolution, fantastique et dans la pratique, le nombre de bénéficiaires concernés va être extrêmement réduit notre collègue a cité à l'instant le chiffre l'impact budgétaire qui chiffre à 20 qui chiffrait à 21 millions d'euros au total et qui devrait concerner au final quelques milliers d'auto-entrepreneurs 6000 pourquoi parce que les autres entrepreneurs dans la pratique, même si leurs chiffres d'affaires pour se même si reçoit pardon des régimes du micro-fiscal micro-sociale augmente, passe de 82000 à 70000 de 32000 270000 euros, dans la pratique, l'effet pratique va être très faible dans la mesure où le seuil de franchise de TVA

Oui, on entend parfois des critiques contre ce PLF en disant qu'on aiderait que les plus riches, les plus gros, le plus important : les gagnants de la mondialisation et inversement, sur les autres, bon, on entend la critique que ce PLF n'aiderait pas assez les les entreprises et et finalement devrait faire davantage, je crois que là on a quand même l'exemple d'une mesure extrêmement intéressante puisque doubler les plafonds du du régime d'imposition des micro-entreprises, c'est simplifier la vie des entrepreneurs c'est ça permet d'aider tout simplement à créer à innover, à entreprendre, je répondrai au rapporteur général que 40 pourcent des entreprises créées depuis le début de l'année. L'ont été sur ce régime de micro-entreprises, c'est donc à un succès du dispositif, parce qu'il permet de fluidifier l'aspect administratif les contraintes et d'avoir une présentation bien sûr, donc moi je pense que ce dispositif cet article 10 et quand même important et qu'il faut le souligner merci beaucoup. Merci, je vais mettre aux voix les 2 amendements de 120 et 564 qui ont reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, ils ne sont pas adoptées. L'amendement 355 rectifier qui le défend. monsieur le président, Monsieur le Ministre, donc c'est un amendement déposé par madame Lamure soutenu et cosignée par de nombreux de nos collègues, alors je ne sais pas si c'est par amour ou par conviction ou par amitié ou par conviction, mais en tout cas c'est un c'est un amendement qui ne qui ne coûtera pas le moindre Euro dans ce budget, c'est, c'est, en effet, simplement un problème de de changement de titre sur l'intitulé de l'article 50 du code général des impôts pour transformer le le le le titre de article en régime micro-fiscal et social en effet madame Namur au travers cet amendement propose de créer un impact psychique auprès des des chefs d'entreprise et de et 2 micro-entreprises puisqu'on était en train de lire que ça ne touchez pas à un nombre important de chefs d'entreprise, c'est peut-être le moyen de les stimuler au travers les propositions qui sont faites dans cet article de de simplification de la fiscalité et des charges sociales qui deviendront forfaitaire et bien sûr, ne plus avoir cet imbroglio de la TVA entre les micro-entreprises et et les entreprises d'aujourd'hui voilà ce en quoi consiste cet amendement. Merci, cher collègue, monsieur le rapporteur de l'avis de la commission. Sur l'amendement 355. l'amendement qui va changer la la face du monde, mais néanmoins seul mérite simplement peut-être de Carrie filer choses quand on dit régime du micro-entrepreneurs des micro- entreprises, ça laisse à penser que c'est à la fois le régime fiscal en entier régime social dès lors qu'il y a pas de relèvement du seuil de TVA, je disais tout à tout à l'heure et que ça concerne uniquement les rejets enlèvement des seuils fiscaux, c'est d'être plus précis, de parler de régime micro-fiscal, donc c'est la raison pour laquelle la commission des finances émis à David sagesse. Merci monsieur le ministre. voilà le compléter peut-être en espérant que le rapporteur général revienne sur son avis défavorable, parce qu'on aura un petit sujet, même si ça a pas d'incidences financières ou un avis défavorable, parce que le régime micro-fiscal qui toucherait que le micro-BIC comme on l'appelle, n'est pas le seul aussi à un seul régime micro-social il y a plusieurs régimes micro fiscaux je ne sais pas si français à cette heure tardive de la matinée, juste, mais il y aurait confusion et je pense confusion qui qui serait à de ce que vous souhaitez, c'est-à-dire pour les entrepreneurs, puisqu'il a, il existe aussi un régime micro-fiscal pour les activités agricoles appelé micro-BA et un autre pour les activités non commerciales, notamment l'activité libérale qu'on appelle micro BMC et donc si on appelle sursis votre amendement changement d'élimination micro-fiscal que celui qui est micro-BIC. Alors que d'autres sont des micro-fiscal sans être dans l'amendement co-présenter alors je crois qu'il y aurait, sorte de de confusion prochaine l'un de vos collègues dira : il faut changer indignation puisque hier, chose de confusion pour l'administration, et pour les entrepreneurs, donc avis défavorable. Avis défavorable, la Commission maintient la vie de sagesse. Donc oui, monsieur Richard pour explication de vote. Pour aller dans le sens du ministre, le code des impôts présente déjà quelques difficultés d'accessibilité et comme membres représentant de Sun à la commission de codification, je ne peux qu'exprimer ma frustration du fait que nous soyons en train de remettre sur l'ouvrage est de clarifier un grand nombre de codes et que le code des impôts ne figure pas au programme, parce que l'administration dont vous relevez donc vous avez donc vous avez la tête Monsieur le Ministre, n'aimait pas particulièrement de bonne volonté, il me semble que le titre dans ce cas-là, est un facteur de confusion endroit si on est titulaire dans un seul chapitre du code des impôts régime micro-fiscal, un régime qui est exclusive des autres alors qu'il y a d'autres régimes micro applicable à d'autres impositions, je pense qu'on. N'amène un risque de confusion supplémentaire, donc il me semble, chers collègues, que tout en comprenant cette idée de donner une qualification cohérente à l'ensemble des dispositions qui concernent les toutes petites entreprises, encadrée par la loi, il vaudrait mieux reporter cette décision. Monsieur le Président ou lourd à la la la volonté de simplifier le code des impôts de madame Lamure mais après consultation des cosignataires nous souhaitons retirer. Donc il est retiré jamais au voir l'article 10 qui est pour l'article 10. Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté. Les article additionnel après l'article 10. Des amendements donc 42 rectifier n'pas soutenu,

la baisse de l'impôt sur les sociétés n'aura aucun impact favorable pour ces entreprises, dans ce contexte, cet amendement vise à remédier à un déséquilibre patents dans la charge fiscale portant sur les petites entreprises, en effet, les bénéfices des entreprises de proximité soumises à l'impôt sur le revenu sont imposés en totalité que ces bénéfices soit utilisée pour rémunérer le chef d'entreprise ou qu'ils soient réinvestis pour accroître les fronts propre à bénéfice égale le chef d'une entreprise individuelle qui doit acquitter des charges sociales, de l'impôt sur le revenu sur l'intégralité du bénéfice qu'ils réalisent légèrement majoritaires qui, juridiquement, sont des travailleurs indépendants sont aujourd'hui les seuls à pouvoir déterminer l'assiette de leurs cotisations alors que le délai, le dirigeant d'une URL d'une SARL d'une SAS imposé à l'impôt sur les sociétés ne subit ces prélèvements que sur sa rémunération, les inégalités, traitement qui en résultent, doivent être prises en compte et réduit autant que possible, c'est donc l'objet de cet amendement, qui propose un mécanisme de suspension de taxation, une partie des bénéfices dans l'entreprise individuelle via un compte d'attente, l'entrepreneur aurait ainsi la possibilité de provisionner ce temporairement et exempt de prélèvements sociaux et d'impôt sur le revenu, à hauteur de 40 pourcent maximum du résultat fiscal de l'exercice.

Donc ces sommes mis en quelque sorte réserve ne serait ni soumis à l'impôt sur le revenu, ni soumis aux prélèvements sociaux. Bon, c'est peut-être. Sur le plan du type d'entreprises individuelles concernés et c'est vrai qu'il ne bénéficient pas de la baisse de l'IS

Par exemple, l'amendement 356 qui propose d'affecter 40 pourcent du résultat annuel, donc au fond multiplie ça par 40 pourcent ça nous fait une assiette potentiel de 43 milliards d'euros, donc voyez que le montant est assez élevé, enfin des vraies valeurs, certes, parfois on parle de d'amendements qui prendre quelques milliers d'euros là on est sur un enjeu potentiel considérable, bien sûr, c'est un peu caricatural ce que je dis, l'ensemble des entrepreneurs ne bénéficieraient pas forcément du dispositif et ne mettrait pas en réserve 40 pourcent dans l'hypothèse où l'amendement

devra avoir un régime fiscal plus adapté le dire, l'un des tueurs dans activité qui est souvent une activité assez fluctuant, les premières années, donc avis demande de retrait pour ces raisons de potentiel risque dans ce public. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le Ministre. Défavorable, donc Monsieur Europe

moi je crois qu'il y a une vraie piste de réflexion, de la même façon que l'amendement précédent, je pense qu'il y a là une volonté d'attirer l'attention des uns et des autres sur la question, bien sûr, on le retire.

Oui, merci Monsieur le Président, donc cet article 10 prévoit de remonter les seuils des micro-bénéfices industriels et commerciaux et des micros bénéfices non commerciaux, et moi j'approuve évidemment cette cette mesure, en revanche, l'article 10 exclus de ce dispositif, les micros bénéfices agricoles, or le système des micro-bénéfices agricoles a été mis en place en 2016 précisément, pour l'aligner sur les 2 autres, et donc je trouve curieux qu'on ait pas associer les micros bénéfices agricoles ce cette augmentation de 2 de ces seuils, d'autant qu'ils sont extrêmement importants, parce que pour tenir compte d'un certain nombre d'aléas climatiques, notamment les micro-bénéfices agricoles, on prend la moyenne des 3 dernières années, donc nous proposons tout simplement par cohérence d'aligner le micro bénéficiaires écoles sur les 2 autres, conformément à ce qui est prévu, dans, dans, dans l'article 10 et nous prévoyons de le mettre en oeuvre, seulement à partir de 1019 pour arriver au terme de cette période triennale en fait 2016, 2019 qui permettra de faire la moyenne sur ces 3 années.

Oui, monsieur le président, mes chers collègues, afin de simplifier la vie des entrepreneurs qu'ils soient artisans, commerçants ou professions libérales et conformément aux engagements du président de la République, l'article 10 du PLF prévoit d'augmenter significativement le plafond de chiffre d'affaires de recettes du régime simplifié pour l'impôt sur le revenu, appelé régime micro-BIC le bénéfice de ce régime conditionné aujourd'hui au respect d'un seuil de chiffre d'affaires ou de recel de 82800 euros l'article 10 du présent projet de loi permet de fixer ce seuil à 170000 dans le secteur agricole, le régime du micro-exploitations dit régime micro-meilleur fonctionne actuellement sur la base du même seuil de chiffre d'affaires de recettes que le régime micro-BIC 82800 parce que, plus que dans tout autre autre secteur, les agriculteurs ont besoin de simplification, sur le plan fiscal, il est proposé à travers de cet amendement d'appliquer l'augmentation du seuil de recettes micro-BIC au seuil de recettes du micro. Merci,

davantage agriculteur de régimes qui ont l'Avantage d'une simplification admnistrative bienvenue pour mais particulièrement chronophage Paris coché cette simplification permettrait l'colonies d'une comptable et donc d'une charge financière. Merci, monsieur le rapporteur de l'avis de la commission. Je ne suis pas certain que ça soit une simple ça simplification comme ça, non, c'est parce que ça a des incidences importantes d'une part sur le montant d'imposition que vous payez des régulateurs et de repart sur leurs droits sociaux pourquoi sur le montant d'imposition, il faut quand on augmente le le le le plafond quand on passe de 80 2800 euros de recettes à 70000 euros lorsqu'on élève le plafond du micro PA, on s'aperçoit que ça peut être défavorable pour un grand nombre d'agriculteurs, pourquoi, parce qu'aujourd'hui, quel est le revenu résultat Net moyen de la branche agricole par exploitation 26809 euros 29 euros c'est le montant moyen et ce montant moyen évidemment par définition, il couvre des des grandes disparités : vous avez beaucoup d'acteurs qui sont

aujourd'hui de 10764 euros à 22110 euros, donc en gros les payer mais ça 4 à 17 euros par mois il peuvent aller jusqu'à 1840 2 euros par mois, donc ça c'est défavorable à un grand nombre d'exploitations qui ont un revenu. être très inférieurs. Donc il se trouverait PDG sur le plan fiscal, sur le plan social ça aussi des incidences, puisque très concrètement ça pourrait priver la MSA de recettes et par définition, les recettes de la NSA, ce sont des droits sociaux pour les agriculteurs, donc la grande disparité de revenus, ça mériterait d'être étudiée, puisque que ça pourrait Célanèse la commission être défavorable tant sur le plan fiscal que sur le plan fiscal, social, pardon à un grand nombre des lutteurs qui bénéficient de revenus beaucoup plus faible que le revenu moyen annoncé. Merci donc avis défavorable. Monsieur le ministre, même avis.

Du micro bénéfice, ça reste un choix volontaire par les aviculteurs il est pas imposée, c'est-à-dire les acteurs peuvent faire ce choix ou un autre choix. Merci donc l'amendement 380 vrai qui fiére est retiré.

du pastoralisme et le plan loup est en cours d'élaboration pour 2010 2023, vous le savez, Monsieur le Sénateur, cependant, c'est un avis défavorable du gouvernement, d'abord parce que tout est privé subventions perçues par les exploitants agricoles se constituent des revenus imposables, c'est un principe général, et lorsque ces aides couvre charges exploitation comme l'entretien des chiens de protection par exemple l'ces frais sont en principe déductible, ces conditions légales d'éligibilité sont bien remplies, la imposition des primes et subventions est alors compensée par l'addition des charges réelles sont censées couvrir lorsque l'aide a pour objet le financement de l'immobilier, l'immobilisation déterminé et bénéficie sur le plan fiscal du régime d'étalement lorsqu'une aide a pour objet de couvrir la perte d'immobilisation et relève du régime des plus-values professionnelles régime qui peut-être très favorable, donc il s'agit ici, monsieur le sénateur, de refuser votre amant parce que votre proposition du rapporteur général en entrée, une différence de traitement injustifiée sur les types d'aides, seules les subventions et prime d'équipement dans le cadre du plan loup seraient exonérées les autres subventions les primes de même nature versés dans d'autres dispositifs demeurerait imposables, et donc une rupture d'égalité : avis défavorable s'il n'y a pas de retrait. Merci monsieur le ministre, donc sur l'amendement 493 rectifier, qui a reçu une demande l'avis du gouvernement de la Commission, un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adoptée. L'amendement 235 monsieur. Monsieur aujourd'hui oui. Merci monsieur le président, Monsieur le ministre, il s'agit d'un amendement de suppression du crédit impôt recherche Seilliere qui représente aujourd'hui 6 milliards d'euros, c'est une une somme énorme et c'est un montant qui a triplé entre 2007 et et 2011 aujourd'hui l'efficacité de ce dispositif sur la recherche n'est pas avéré et nous attendons du gouvernement qui nous prouve le contraire, jusqu'à présent, nous n'avons pas vu ses arguments pire pour 6 milliards, on constate que la France continue de chuter dans le dans le classement sur la recherche et développement, pourquoi essentiellement parce que le le c'est hier profite aux grands groupes industriels qui l'utilisent comme un outil d'optimisation fiscale on a finalement instauré chez nous un petit, un petit paradis fiscal de de 6 milliards d'euros, le recours que font ces grands groupes, à la recherche et développement par des stratégies internationales pour lesquels les fessées hier ne représente qu'un moindre un moindre intérêt je voudrais juste citer l'exemple d'Airbus qui touche énormément de Seilliere et qui a fermé son centre de recherche et développement

je voudrais juste évoquer une injustice terrible alors que l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, un taux d'échec de 90 pourcent c'est-à-dire que malgré

par ailleurs, je voudrais finir par un un point sur l'organisation budgétaire le CRC une boîte noire, c'est-à-dire que c'est un un instrument dans lequel nous perdons 6 milliards de recettes fiscales conclure je finis et sur lequel le Parlement n'a aucun pouvoir pour mesurer la réalité des engagements qui sont faits dans le domaine de la recherche, Jean merci.

à Toulouse justement chez Airbus et nous avions rencontré un grand nombre de sous-traitants de 1er de second rang qui bénéficiait du crédit impôt recherche et et et ce qu'il était ressorti, c'est qu'ils étaient présents en France, il y avait notamment des entreprises allemandes sous traitant des et d'un bus et pourquoi il n'était pas en Allemagne, pays qui produit beaucoup d'ingénieurs étaient précisément en France car ils bénéficiaient du dispositif du crédit d'impôt recherche donc je pense que c'était un des rares régime fiscal sur lequel la France se distingue vraiment par un Avantage compétitif extrêmement important ça coup élevé c'est vrai ça, quoi rêver, ce n'est pas parfait, il y a sans doute, comme partout, des abus, même s'il y a une expertise ce est descendue parfois des effets d'aubaine, ça n'empêche pas, c'était 10 à la de refinancement de recherche mais l'analyse de la Commission, c'est que sur le nous aurions encore moins de recherche privée en France et nous savons aujourd'hui quand on regarde les chiffres, déchets et du commerce extérieur, que là où la France de lutter, c'est pas uniquement par rapport à par des pays qui ont des coups bas par des avancées technologiques, pas de la montée en puissance mots tu regardes ceux qui décident de la recherche et la recherche appliquée, notamment dans les entreprises, donc évidemment avis défavorable sur cet amendement.

monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le groupe de de l'Union centriste ne peut pas ne peut pas laisser dire dans cet hémicycle que l'intérêt du crédit impôt recherche n'est pas avéré comme je viens de l'entendre à l'instant, j'ai aussi fait partie de la commission d'enquête qui est cité dans les oeufs, la motivation de de cet amendement et de cette commission d'enquête partout, j'ai entendu dire de la part des entrepreneurs combien il pouvait s'appuyer sur le crédit impôt recherche pour leur développement et on sait bien que les conditions de la compétitivité de nos entreprises françaises est lié à leur capacité d'évolution et je ne vois pas comment demain il pourrait encore y avoir des travailleurs en France si les entreprises ne sont pas compétitives au plan national et international, et donc si elle n'innove pas, aujourd'hui, on est dans un monde où les choses bougent beaucoup, on le voit bien avec le développement du numérique et donc imaginer que tout cela puisse se faire sans l'innovation me paraît totalement surréaliste, donc il y a un impératif d'améliorer la compétitivité des entreprises françaises, le crédit en optant impôt-recherche est vraiment l'un des outils enviée dans le monde entier à la France, pour cela, donc ne nous séparons pas de cet outil, qui en plus permet de recruter dans dans des entreprises, des chercheurs de haut niveau et n'oublions pas comprendre l'Europe de nous sommes engagés dans ce qu'on appelle la stratégie de Lisbonne en en 2000 vers le fait de consacrer 3 pourcent de notre produit intérieur brut à la recherche, dont les 2 tiers par les entreprises et nous en sommes là encore donc, il faudrait au contraire que les entreprises recourent encore beaucoup plus au crédit impôt recherche, c'est-à-dire développe considérablement leurs efforts de recherche pour que demain nous puissions à la fois résoudre la question de l'emploi qui est absolument crucial dans notre pays, la question des exportations, enfin de la balance commerciale permet je l'évoquais tout à l'heure et je dirais une bonne santé de nos entreprises. Et Madame Bruni pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président, oui au contraire de de mon collègue, moi j'ai dit, effectivement, ça ça bénéficie à des grosses entreprises mais ça bénéficie aussi beaucoup à des plus petites entreprises moi chez moi ça bénéficie à certaines petites petites entreprises du textile, il nous en reste encore un petit peu et sincèrement il nous voir souvent en disant : surtout qu'on puisse conserver, en fait, ce dispositif et ce dispositif sincèrement c'est pas 3 lignes sur une feuille de papier administrativement justement c'est c'est très lourd quand des entreprises, elle le demande, je peux vous dire quelle qu'elles y passe du temps, après un moment donné il y a eu justement beaucoup de contrôles fiscaux qui ont été déclenchées par la demande de crédit d'impôt, je pense qu'aujourd'hui c'est : c'est beaucoup plus serein, donc c'est franchement, ça a été, c'est encadré c'est surveillé, c'est un dispositif dont on a besoin et puis moi je vais vous dire aussi en entreprise, on parle d'investissements, les investissements, ça représente toujours un coût, donc comme ici avec le crédit d'impôt recherche en revanche, on a un retour sur investissement et c'est ça qu'il faut regarder et dans ce retour sur investissement sont des entreprises et encore des emplois en France, vous pleurez parce que il y a pas d'emploi et vous voulez les détruire quand on a des bons dispositifs c'est vraiment scandaleux, moi ce que j'ai pu entendant dans votre intervention. Si Madame Goulet pour explication de vote. Oui, Monsieur le le président et ses Ministre, mes chers collègues, moi je, je ne doute pas qu'on ait besoin de d'investissement. Bon, aujourd'hui, pour la recherche, j'ai lu le le rapport de notre de notre Sénat sur le crédit impôt recherche et je sais les critiques qui sont faites et j'entends aussi les les points positifs mais je voudrais aussi relevé dans dans dans l'intervention de notre collègue du groupe communiste républicain citoyen est désormais écologique. Le lien et la corrélation entre un certain nombre d'aides et des licenciements, et vous pourrez pas franchement déconnecté ces ces 2 éléments, en sachant que que les licenciements boursiers, pose aussi un certain nombre de problèmes et que des entreprises qui reçoivent des subventions à un titre ou à un autre dans un, dans le même temps, procèdent à des licenciements, moi je suis dans un département où on a eu dans le temps, Moulinex avec un certain nombre de licenciements posthume avec beaucoup de subventions et parallèlement toutes un nombre extrêmement important de licenciements, donc oui le crédit impôt recherche, c'est nécessaire, et celle des petites et moyennes entreprises, hé oui, il y a un problème quand des entreprises touchent des sommes importantes au titre du crédit du du crédit impôt recherche et qu'en même temps il licencie du personnel, donc à la fois, il faut le garder et en même temps peut-être qu'il qu'il faudrait donner un peu plus de 2 conditions de maintien de l'emploi aux entreprises qui pourraient en bénéficier, je pense que ce serait pas scandaleux. le financement de la recherche, fut-elle privée sur des crédits de l'État, bien au contraire même, bien au contraire, mais là ce que nous constatons, c'est que ces 6 milliards, ils ne vont pas, ils ne vont pas la recherche premièrement vous nous citez les PME aujourd'hui, c'est celle qui le touche le moins l'essentiel des 6 milliards sont captées par les grands groupes industriels avec une politique, je l'ai dit d'optimisation fiscale qui n'a rien à voir avec la recherche sur la réalité de ce qui se passe dans le monde de la recherche, on constate que les 6 milliards que nous avons dépensé ont eu aucune influence sur la précarisation majeur des chercheurs de plus en plus importante et que, par ailleurs, le nombre de docteurs à diminuer, nombre de docteurs a diminué donc c'est un échec, il faut le reconnaître, qu'il faut trouver d'autres dispositifs et les dispositifs qui sont mis ailleurs en Europe, sont sains du point de vue des principes et de la morale, je pense à l'Allemagne, ce sont les subventions sur projet il y a un projet, enfin un appel d'offres, on regarde les dossiers et en finance et on peut constater si le résultat de la recherche et équivalent et équivalent à ce qu'on a financé la encore une fois, c'est 6 milliards c'est une boîte noire, nous mettons de l'argent dedans et nous ne savons pas ce qu'il ce qu'il devient. Merci, cher collègue Monsieur Reina le pot, explications de vote. moi je trouve que dans dans ce qui vient d'être dit, il y a un peu de de vérité partout les l'essentiel étant de, de, de, de garder la raison à la fois dans la critique, il y a toujours des éléments de cette nature des sujets bien sûr, il y a forcément toujours des. Les entreprises qui utilisent la mauvaise gestion, si je puis dire, le crédit impôt recherche et en même temps il y a un dispositif qui globalement utile et je crois que ça aussi il faut le il faut le partager, mais moi j'ai tendance à dire aussi que le crédit d'impôt recherche et il faut le regarder dans un ensemble qui est la fiscalité de l'entreprise et que d'une certaine façon le crédit d'impôt recherche, il a permis aussi finalement 2 d'améliorer au sens des entreprises, la fiscalité et de la rendre plus compétitive, notre fiscalité par rapport à 10 implantations qu'on va choisir des grandes entreprises et quand elle choisit choisissait la France elle, regardez le taux d'imposition mais le regarder aussi le crédit d'impôt recherche c'est sur une globalité que les choix des entreprises en tout cas des grandes entreprises se se réalise et donc le sujet peut être revu en tout cas dans ces montants au moment où nous aurons baissé le niveau d'imposition globale des entreprises, je crois que c'est comme ça aussi qu'il faut qu'il faut regarder, regarder les choses mais en même temps l'idée de dire que l'on soutient finalement on en a parlé hier et avant hier l'amélioration pourquoi donc je crois hors charges et hors coûts je trouve que c'est très important et donc effectivement le crédit impôt recherche, pour l'instant, a toute sa place dans ce dispositif global, je crois que, au fur à mesure du temps, il pourra peut-être être réajustés en particulier lorsque nous aurions, nous aurons une fiscalité générale l'entreprise dans la moyenne européenne, c'est un élément important du de la réflexion, me semble-t-il.

je me suis quand même fait une une bonne idée de ce que ça représentait, moi je sais que le groupe CRC, tout comme nous, et est attaché à l'emploi, et s'il y a bien, dans les évaluations qui ont été faites du crédit impôt recherche depuis qu'il a été réformé en en 2008, il y a bien un point qui est ressorti, c'est qu'il a été favorable à l'emploi, peut-être pas au nombre de brevets déposés, mais au moins, au moins à l'emploi sur les brevets déposés vous dit que, effectivement, il y a des modèles différents en Allemagne sur appel à projet ou autres, oui, mais chez nous, c'est un petit peu pareil, notamment avec la je pense la la réforme à venir de l'ANR on on souhaite des crédits ont été abondé sur ce budget, c'est pour ça que, on l'a salué, au niveau de la Commission,

le crédit impôt recherche est quelque chose qui fonctionne certes, c'est 90 pourcent des dépenses fiscales de la mission, mais c'est quelque chose qui, qui fonctionne et qu'il faut encourager,

Le crédit d'impôt recherche un dispositif qui fonctionne, qui marche et je crois qu'il faut faire attention quand on y touche, porter atteinte, en concurrence avec des pays qui ont accéléré sur la recherche, je pense à la Chine par exemple, et si on veut perdre des places, la meilleure façon, chers amis, se serait notamment de s'en prendre au crédit d'impôt recherche ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet d'aubaine qu'il ne faut pas le contrôler ou l'évaluer, il y a d'ailleurs eu une proposition à l'Assemblée nationale autour d'Amélie de Montchalin sur la question notamment du nombre de doctorants recruter, c'est un, c'est volonté de travailler avec les premiers concernés qui sont les chefs d'entreprise pour évidemment améliorer par exemple un certain nombre de contrôles de conditions, on peut réfléchir à des éléments comme le verdissement supplémentaire du crédit d'impôt recherche on peut continuer à travailler sur le contrôle des effets d'aubaine, mais je crois qu'il faut être extrêmement prudent face à un mécanisme qui a fait ses preuves, c'est dommage de Detrick de vouloir détricoter ce qui fonctionne bien, merci beaucoup. Merci, cher collègue Monsieur Capo-Canellas pour explications de vote. Oui, merci Monsieur le Président, mais déjà Collet, simplement je vais passer un message, c'est que je crois que dans ces matières-là lorsqu'il s'agit à la fois fiscalité d'attractivité des entreprises, on doit avoir pour règle de garder une certaine stabilité, une lisibilité des dispositifs et le crédit impôt recherche est des dispositifs et il y en a pas tant qui du point de vue mondial nous identifie comme étant un pays qui est attractif et qui souhaitent développer indécent de recherche je crois qu'il y a eu des effets parfois un peu, au contraire, ça peut arriver, l'ensemble des dispositifs mais il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et que ce dispositif a en tout cas permis aussi à des entreprises françaises de garder, de développer leurs centres de recherche dans notre dans notre pays et ça ça donc du sens. Merci Michel, collègues, donc je vais mettre aux voix l'amendement 235. Pardon. Ce qui a pu pour explication de vote si ça peut être aussi. Oui, il y avait une explication de vote, monsieur le président. Très rapide. Notre industrie vieillissante, on est dans une concurrence mondiale de plus en plus effréné avec l'Asie, qui est de plus en plus efficaces et qui développe sa recherche notre arme principale, ce sont nos cerveaux et ce, c'est la recherche et le développement, si on ne met pas le paquet sur la recherche et le développement à travers, comme l'a dit monsieur notamment l'attractivité de nos industries, nous sommes condamnés. Sinon à disparaître, je ne voudrais pas paraître pessimiste mais a décliné, c'est totalement aberrant de vouloir supprimer les dispositifs qui permettent à la fois l'innovation en France et l'attractivité de notre territoire. jamais au voile l'amendement 235 qui a reçu un un double avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adoptée. Je mais au voilà recycle 10 bis qui est pour. Qui est contre.

déjà faible des zones rurales épais rural constitue un point d'appui indispensable de la réalité revitalisation rurale espérer, c'est pourquoi il est proposé d'inclure les sa neutralité du département où la population était à 30 habitants par Timothée carré, soit les 7 départements les plus ruraux et le second amendement que je défends même temps proposé ne permettant plus large les départements où la population était ailleurs, à 35 habitants au kilomètre carré, c'est qu'nous reste bon à 14 départements. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur, l'avis de la commission.

n'étaient pas toujours satisfaisantes et je le dis clairement, à nouveau, elle est partie, roman à satisfaisante lorsqu'il s'agit des collectifs budgétaires et en 2015 dans le cadre du projet de loi de finances active, il faut 2015 nous avions examiné dans une extrême urgence les les réformes du zonage des aides RER sans avoir à la et d'avoir un vrai débat de fond sur cette question du zonage qui pose des difficultés et c'est la raison pour laquelle il y a sans doute des amendements donc encore une fois, je reconnais volontiers que ce zonage n'est pas parfait que ce zonage a été adopté dans le cadre d'une loi de finances rectificative, celle de 2015, qui a été examinée dans les conditions non satisfaisante que je signalais et je rappelle et sur le fond, je partage ce que dit Jean-Claude Requier bon néanmoins cet amendement pose une difficulté, c'est que vous le lisez. Il est malheureusement. Non, ce précis et il veut pas tourner quand on vous dit les centralité,

Même vote. Même donc il n'est pas adoptée. Donc, nous passons à l'article Dister un amendement 610 du gouvernement, monsieur le Ministre bienvenue donc je vous passe la parole sur cet amendement 610. Merci monsieur le président, monsieur le rapporteur général, monsieur le président de la commission des finances d'abord avoir le plaisir de vous présenter la nouvelle secrétaire d'État. Qui va siéger dès cet après-midi au banc, l'amendement qui vous est présenté et tu un amendement de coordination visant la fusion des différents régimes de recettes commerciales accessoires réalisés par les exploitants agricoles rattaché au bénéfice agricole. Si Monsieur le Ministre, donc avis de la commission.

Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté. Après l'article Dister sur les articles additionnels monsieur rapporteur Vouziers, prendre la parole. Nous avons un très grand nombre d'amendements en discussion commune, nous avons 7 qui vise à réformer la déduction pour pour aller à il s'agit, discussion important de façon à peut-être rendre notre discussion plus compréhensible vous expliquer un petit peu la position de la commission des finances, donc je disais 4 amendements, discussions communes, il s'agit tout simplement de réformer le régime de la direction pour aller à et sans doute de progresser vers une meilleure contribution à la fiscalité agricole la stabilisation du revenu des entreprises du secteur, vous savez que celle-ci est mise à mal par la coterie qui était station d'une large gamme de risque sont particules activités agricoles, c'est la volatilité des prix, c'est l'Exposition à des aléas climatiques, c'est aussi les risques sanitaires, bref, nous avons à cet homme d'aléas et c'est précisément pour ça qu'il a un régime de la direction pour aller la fiscalité agricole, vous le savez, comporte plusieurs dispositifs spécifiques qui permettent sans doute, mais insuffisamment de compenser les effets de ces aléas et nous avons examiné à l'instant, la déduction pour aléa que les amendements, discussions entendent améliorer pour certains d'entre eux, il y en a d'autres qui veulent laisser sublimer en quelque sorte puisqu'il va aller jusqu'à instaurer un dispositif de taux assurance fondée sur la constitution d'une épargne de précaution, bref tous ces amendements vont dans le bon sens sans doute. Et. Je remarque qu'ils viennent de différents groupes qui se rallient, en tous les cas, tout ça, une idée commune, celle qu'il faut réformer le dispositif, donc c'est la raison pour laquelle la commission des Finances voit plutôt d'un bon oeil ces amendements, il faut en effet reconnaître que la baisse de la valeur ajoutée par actif agricole, celle-ci a baissé de plus de 12 pourcent 2016, a de quoi nous alerter, d'autant plus que face à la volatilité des cours et des revenus agricoles, les impôts sur le revenu, apparaissent moins élastique, même s'ils sont par la réflexion, légèrement, même s'ils donc il est donc plus que justifié d'avancer vers une fiscalité quel qu'ils soit plus protectrice qu'elle ne l'est aujourd'hui, et par conséquent il faut sans doute franchir le pas vers un soutien de la fiscalité directe à l'école et l'effort d'épargne de précaution que souhaite entreprend les entreprises de la branche, cela est d'autant plus nécessaire que les interventions en crédit, tu as signé internationale qu'il faudra renforcer son mal provisionnés par les Budgets, écoles et c'est ce budget budgétisation non pas seulement pour effet d'affecter la sincérité budgétaire mais aussi ils installent parfois un climat anxiogène pour les acteurs du secteur, j'ai donc dit la diversité des États, des amendements, amendements, tous les bons donc cela témoigne sans doute d'une volonté consensuelle de réformer les choses, donc on ce contexte, il faut cependant toutefois tenir compte de la diversité des dispositifs proposés qui se distingue sur telle ou telle point certains vont vers le calcul de la réserve de précaution d'autres réformes, les conditions d'emploi donc les conditions de réintégration résultat et c'est la raison pour laquelle, vous comprenez que ces amendements, même s'ils vont tous dans le même sens, se révèle complexe. Et. Nous devons légiférer sans nous tromper ça nécessite un travail d'instruction qui soient, soient mieux et il est difficile de l'entreprendre, à l'occasion de l'examen d'moment de séance c'est vrai que nous avons largement avancée au Sénat, dans lequel les travaux réalisés pour améliorer la compétitivité de traîner, culture et vous vous souvenez de la proposition de loi qui avait été porté au Sénat sur la compétitivité, c'était culture l'article 6 comportait à dispositif remarquable, une avancée à mon sens, on la retrouve d'ailleurs dans un certain nombre d'amendements néanmoins tout est perfectible. Et. J'ai vu que lors des débats du PLF à l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, vous aviez pris un engagement, vous avez peut-être réitérer à l'instant un engagement ferme de réformer en profondeur la fiscalité agricole en associant à cette préparation de cette réforme, les parlementaires intéressés je c'est la raison pour laquelle tout homme ralliant à la démarche des différents acteurs d'amendements, je disais bien de tous les bancs, il y en éprouvant parfois plus de sympathie pour certains amendements que pour d'autres, je demanderai leur retrait décemment si bien entendu et je me réjouis que le ministre arrive à l'instant, si bien entendu, Bruno Le Maire, si le ministre ne confirme son intention de réformer en profondeur cette fiscalité et tient devant la Haute rassembler les engagements qu'il a pris dans l'Assemblée nationale et dans ce cas là, je le retrait et, bien sûr, avec également l'intention réaffirmée par un certain nombre de membres, mais en tout cas pour ma part de travail avec voudrait que le gouvernement a une réforme pour vous donner cette fiscalité, il faut en effet trouvé un régime satisfaisant face à des volatilité des cours qui sont de plus en plus nombreux pour les raisons que j'évoquais à l'instant donc voilà c'est un petit peu parce que je vais vous dire avant que nous examinions c'est article et que j'entends le ministre. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre vous souhaitez apporter une précision.

donc il y a des différentes pole-position pour être ministre, on peut avoir voté contre le budget on peut être en dehors d'avis politique, on peut avoir été plus budget voilà en tout cas de maman et la D avoir le plaisir de travailler avec elle, tout à l'heure. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre. Moi, je suis heureux de constater que le rapporteur général est revenu en pleine forme. Cela me réjouit, je voudrais lui confirmer que je suis prêt à ouvrir le débat sur la fiscalité agricole et davantage que prêts, nous avons commencé les travaux nous avons commencé à consulter les organisations syndicales et avec Stéphane Travert, le ministre de l'agriculture nous voulons ouvrir ce chantier-là. Chacun sait que la fiscalité agricole aujourd'hui n'est pas satisfaisante qu'peut être amélioré, chacun voit bien que face à la volatilité des prix agricoles, il y a besoin d'offrir de nouveaux instruments aux agriculteurs, que ce soit face aux aléas climatiques renversement de tendance à l'effondrement des prix, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur du port avec un effondrement à nouveau des cours du porc qui pose des problèmes absolument majeur à nos producteurs et à nos agriculteurs, il faut impérativement avoir des dispositifs efficaces en matière de fiscalité pour soutenir nos producteurs. En revanche, sur les propositions qui sont faites dans l'amendement, moi il me semble que ça n'est pas les solutions adéquates pour nos agriculteurs le plafond global de déduction qui est fixé à 27 pile : Euro : je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le modifier et de l'élever davantage ça coup important pour les finances publiques et je ne suis pas certain que ça corresponde vraiment à la demande des agriculteurs sur l'aléa économiques. Vous avez retenu comme définition de l'air économique et une baisse de la valeur ajoutée égale à 5 pourcent de la valeur moyenne des 3 ou 5 ou dernière exercice une baisse la valeur ajoutée en moyenne de 5 pourcent ça correspond à ce qu'est la réalité économique courante d'un agriculteur et producteur industriel ou de quelqu'un qui travaille dans les services, il me semble pas qu'on est dans l'aléa, on est dans la réalité économique et par ailleurs on voit bien que les effondrements de prix agricoles peuvent être beaucoup plus brutaux que simplement 5 pourcent hélas. S'agissant de l'utilisation de l'AD-PA pour l'équitation d'immobilisation, moi, je vous rappelle que la réforme qui avait été conduite en 2012, la déduction pour investissement mais supprimer cette possibilité d'utilisation pour l'acquisition d'immobilisation et moi je suis alors je vous le dis très sincèrement extrêmement sceptique sur l'idée de revenir là-dessus parce que ça incite nos agriculteurs à acheter des matériels dont ils n'ont pas nécessairement besoin qui ensuite vont peser sur le compte d'exploitation et sur la rentabilité des exploitations donc tout ça pour vous dire que je rejoins la position du rapporteur général, je vous suggère de retirer cet amendement, je confirme mon engagement, l'ensemble des amendements sur ce sujet-là, je confirme mon engagement d'ouvrir la réflexion soit fiscalité agricole et que le ministre agriculture Stéphane Travert pour répondre aux préoccupations légitimes les producteurs. Monsieur le ministre, donc je m'adresse aux signataires des des amendements qui sont en discussion, commune de 397 rectifier 400 de rectifier 526 rectifier 582 403 rectifier 519 est-ce que vous êtes d'accord pour retirer ses amendements, monsieur, d'abord, le 397 rectifier monsieur Delcros. Oui, oui je contenu de, de, de ce que des engagements pris par le ministre sur une reprise de la fiscalité agricole qui a effectivement besoin d'être mis à faire, je retire cette amendement.

moi je lis que j'avais fait un rapport avec Monsieur Bizet, commission des affaires européennes, on a vraiment engagé déjà une réflexion, donc moi je vais vous dire très bien pour faire des réflexions, on n'arrête pas de nous en parler depuis le PLFSS sur un tas d'chantier que vous allez mettre sur la table, seulement un chantier, il faut à un moment donné que ça se termine et les agriculteurs, ils n'en peuvent plus d'attendre et les crises malheureusement avant on pensait que c'était une fois de temps en temps, une fois tous les 10 ans, aujourd'hui elle devienne pérenne, il y a pas de réponse, donc on les retire, on vous fait confiance, mais sincèrement, la réponse c'est pas dans 3 ans, c'est pas 2020, 2025 c'est 2000 18 heures 30 juin 2018 au plus tard, on a trouvé une solution et une réponse pour nos agriculteurs qui attendent vraiment ça merci.

Madame Voynet et retirée aussi écoutez donc les 7 amendements sont retirés. Et nous passons à l'article 10 squatter des amendements de la commission, le sens de monsieur le rapporteur.

donc, nous passons à l'agriculture, au logement et donc cette amendement numéro 102. Pour objet tant le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés pour les plus-values dégagées lors de la cession de locaux professionnels ou encore des terrains à bâtir, en vue de la construction lorsque le cessionnaire du site civils bénéficiant du régime de l'article 239 dans une société civile ayant posé à la construction en vue de la vente, donc c'est une ouverture qui permettrait au cessionnaire de bénéficier du régime incitatif pour faciliter la concrétisation de passion, de transformation de locaux professionnels en logements, donc c'est ça l'objet voire plus. De locaux professionnels transformés en logements et c'est l'objet de l'art de l'amendement 102. Et monsieur le rapporteur, monsieur le Ministre, l'avis du gouvernement. D'abord je voudrais remercier les sénateurs pour leur compréhension sur la fiscalité agricole même il a très bien dit, c'est un sujet absolument majeur, je pense avoir particulièrement conscience des attentes des agriculteurs sur ce sujet, donc j'ai pris un engagement et il sera tenu sur l'amendement proposé par le rapporteur général, je crois qu'il va dans le bon sens, ça permet de répondre aux besoins de logements dans les zones tendues donc comme ça va dans le bon sens, c'est un avis favorable. Merci, Monsieur le Ministre,

Prima. Merci Monsieur le Président, les dispositions de l'article 212 du Code général des impôts mettent donc à l'impôt sur les sociétés autorégule de 19 pourcent les plus-values nettes résultant de la cession d'un local à usage de bureaux ou à usage commercial à condition que l'acheteur l'acheteur locaux en logements dans un délai de 4 ans, en pratique, ce délai de 4 ans peut être un peu juste, puisque vous connaissez les difficultés à transformer les choses rapidement dans ce pays et donc afin de rendre possible cette cette transformation, nous souhaitons passer ce délai à 6 ans. Merci, monsieur le rapporteur général avec la Commission. Un sujet qui est déjà connue puisque la dernière nous avions étendu le délai qui a été cité à l'instant de 3 ans à 4 ans.

d'impôt sur les sociétés, faut-il pour autant le passé à 6 ans ça paru un petit peu et de la Commission, et donc on souhaite rester l'état de ce qui a été votée, Asnières, c'est-à-dire 4 ans après l'extension, je dirais, de 3, 4 ans, donc une demande de retrait pour cette raison. Merci monsieur ministre. Même avis que le rapporteur, j'ajoute, si ça peut vous inciter au retrait que le texte prévoit déjà dans certaines situations, un délai de transformation supérieure à 4 ans donc, soit retrait soit avis défavorable.

Oui Monsieur Prix monsieur, madame la ministre, mais cher collègue, l'article 10 secrétaire donc dont inciter les entreprises à vendre des terrains, des locaux commerciaux et des bureaux pour créer des logements, il prévoit donc jusqu'au 31 décembre 2020 l'retour réduit d'impôt sur les sociétés de 19 pourcent des plus values réalisées lors de ces sessions sous condition d'un engagement de construction de transformation des biens vendus en logements dans un délai de 4 ans notre amendement Vendôme, nous semble-t-il, dans le sens des ambitions du gouvernement et propose d'étendre l'application du taux de 19 pourcent sur les plus-values réalisées par les organismes HLM, notamment à l'occasion de vente de locaux commerciaux ou à usage activité située en rez de chaussée des immeubles à condition bien entendu que ces plus-values, soit réinvesti dans un délai de 4 ans dans la construction, l'acquisition ou la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs sociaux, cette mesure est d'autant plus importante que les organismes HLM sont de plus en plus incités à céder des locaux dans le cadre de diverses opérations de restructuration. L'avis de la Commission, monsieur le rapporteur. La portée de cet amendement assez réduit, vous ça ne concernerait que les seules activités. où les bailleurs. Ne serait pas exonérés d'impôt sur les sociétés, mais la, la, véritables raisons du, de l'avis défavorable de la commission, c'est plutôt la difficulté qu'il y a contre les applications du dispositif, comment peut-on vérifier que le bailleur social dans le délai de 4 ans a réinvesti les sommes véritablement revisiter les sommes donc un vrai problème de suivi et dispute, il n'est pas paru évi opérant, c'est la raison pour laquelle la Commission était défavorable.

Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté, même vote pour le disque inquiets. Un vote à l'article 10, sexe, yes, je suis saisi d'un amendement de 174 rectifier bis c'est Monsieur Lefebvre, qui le défend. Oui, Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, sur la base d'un rapport parlementaire, en date du 8 octobre 2014 le gouvernement précédent avait fait adopter l'art une réforme des zones de revitalisation rurale désormais quelques l'intercommunale de critères ont été retenus pour définir une ZR1 une densité de population et le revenu par habitant n'est plus non plus compte du critère dit de très faible dans le temps, cité pardon, ces nouveaux critères ont entraîné des conséquences très dommageable pour de nombreux territoires ruraux en effet un certain nombre de communes rurales ont perdu leur classement alors que le regard extérieur STIC n'ont pas changé si l'amendement adopté à l'Assemblée nationale, initiative du gouvernement va dans le bon sens maintient notamment à titre provisoire, jusqu'au 31 décembre 2019 du dispositif du dispositif des intérêts aux communes qui en sont sortis et qui ne sont pas couverts par la loi montagne de 2016, il met en avant des erreurs de la réforme, toutefois, il importe de se poser la question suivante : que va-t-il se passer après cette période de transition au 1er janvier 2020, cette interrogation amène l'auteur de l'amendement voir ici qu'une mesure palliative en effet rien exclu un nouveau prolongement lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2019 afin d'éviter que chaque année, devienne une année de doutes pour de nombreux élus locaux et les proposer de rétablir des critères de classement des communes situées en EDF, tels qu'ils existaient avant l'adoption de la loi de finances actif il captive de décembre 2015 on est bien conscient que le rétablissement des anciens critères poseront un certain nombre de problèmes de PC qui jouissent de bénéfices du nouveau zonage toutefois à préciser que les anciens critères posés beaucoup moins de problèmes que ceux d'aujourd'hui, l'amendement du gouvernement illustre d'ailleurs bien ce jugement avant merci. Merci l'avis de la Commission, monsieur rapporteur général. dans la précipitation dans la finance rectificative avec une difficulté d'absence d'expertise et et donc Los aurait mérité un meilleur débat néanmoins je pense que l'amendement que nous venons d'examiner n'est pas, ne règle pas tout puisqu'il concrètement au régime antérieur à cette réforme de la loi de finances rectificative pour 2015, cette solution aurait des inconvénients importants, je crois d'ailleurs l'auteur de l'amendement, histoire d'amendements sont conscients puisque nous a dit qu'à la fin, je lis l'auteur de l'amendement est conscient que le rétablissement de critère posera de problèmes aux communes et aux PC, PC Kiber jouissent du bénéfice du nouveau zonage très concrètement ça aboutirait à faire sortir 3600 communes du nouveau zonage, donc vous imaginez les difficultés d'application pratique, donc il a paru à l'État la commission qu'il valait mieux se donner un petit peu de temps avant de prendre des décisions qui aurait des conséquences aussi importante, donc demande de retrait sinon avis défavorable. Et Monsieur le Ministre. Oui, même avis que le rapporteur général, monsieur le président, c'est un sujet les derrière qui est absolument majeur pour chacun d'entre nous ici que connaît bien Christophe Castaner, je rappelle juste que nous avons décidé du principe d'une réforme des aides RR en 2015 dans le prolongement d'une mission parlementaire eu des travaux tout à fait remarquables qui ont été faits, aussi bien par le Sénat, que par l'Assemblée nationale, cette réforme a été prévue en et les faire est entré en vigueur au 1er juillet 2017, donc nous avons désormais des nouveaux critères de classement que vous avez rappelées qui tient compte de la densité de population pour créer une logique de développement économique, de projets, nous avons par ailleurs en première lecture de la loi de finances pour 2018 instauré à l'Assemblée nationale à l'article 10 sexy qui prévoit le maintien en ZR jusqu'au 31 décembre 2019 de toutes les communes qui sont sortis du classement au 1er juillet 2017, donc on a fait cette prolongation, justement pour éviter qu'il y a une rupture et que ce soit trop brutal pour ces communes donc revenir en arrière, va créer des difficultés considérables parce que celles qui se trouvent maintenu vont avoir des interrogations, ceux qui sont sortis, voire des interrogations aussi, donc j'ai peur que ça crée beaucoup de confusion et beaucoup d'insatisfaction, enfin, je rappelle que nous nous sommes engagés avec l'ensemble du gouvernement, avoir un rapport sur la mise en oeuvre la sortie progressive du dispositif des et derrière pour les communes qui ne répondent plus aux critères parce que bien entendu, je comprends parfaitement leur inquiétude, c'est normal qu'on évalue les conséquences sur ces communes donc ma recommandation cette un retrait sinon avis défavorable. Merci monsieur le ministre, donc 2 demandes de retrait ou sinon avis défavorable, j'ai eu des explications de vote Madame Goulet. monsieur le président, Monsieur le ministre, le rapporteur général a très bien dit, c'est une une réforme qui est le le le modèle de de ce qu'il faut pas faire, bien qu'il a eu un rapport parlementaire, les territoires ont besoin de lisibilité et ils ont aussi besoin de de sécurité en même temps, ce sont les derniers qu'on écoute quand il s'agit de de modifier ce type de ce type alors moi je, je suis très ennuyée parce qu'à la fois je comprends très bien les inconvénients de l'amendement et en même temps, il faut faire. Quelque chose alors Monsieur ministre vous qui avait été ministre de l'Agriculture, Économie, qui connaissez si bien les territoires il faut il faut nous proposer quelque chose, soit des préfectures bienveillante soit remonté les difficultés qui arrive, commune par commune, nous, territoire par

pour les mêmes territoires donc à la fois on peut pas recommencer, on peut pas défaire d'une façon erratique ce qu'on a fait d'une façon erratique parce que du coup, on va se retrouver avec 2 erreurs de procédure en même temps, celle qui l'a instaurée, celle qui voudrait la mettre en marche arrière, donc on a un problème de procédure et en même temps on a un problème de fond, donc là aussi monsieur ministre il faut nous aider à trouver une solution qui permette de répondre aux besoins des territoires qui sont nombreux, parce que l'amendement provient vraiment du d'une d'une d'un besoin des territoires, donc il faut trouver l'adéquation entre la demande et la procédure adéquate, c'est : c'est l'équation à laquelle nous sommes soumis me ce matin donc, l'amendement est légitime sa solution de l'pas, il faut qu'on en trouve une. Et monsieur Gagnier pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur Islam, messieurs les ministres, le Ministre. Je pense que nous allons très certainement un vers un retrait de cet amendement, toutefois, je voudrais en profiter quand même pour évoquer les les causes profondes de la nomme à vie qu'il présente. Car en réalité ce qu'on cherche à avoir avec les zones de réislamisation rural c'est le caractériser, quelque part, ces territoires en déclin, ces territoires en perte de vitesse, etc, et la problématique qu'il y a et qu'effectivement on n'a pas assez examiné, c'est qu'on a voulu introduire ce qu'on appelle la valeur médiane, il faut à cet égard, je voudrais quand même dire que il faut faire très attention dans ce domaine où la mathématique se mêle à la fiscalité parce que la valeur médiane, tout le monde la considère comme la la la Pierre philosophale mais en réalité, je peux vous citer un exemple très, très concret ou de territoire avec le monde, même nombre d'habitants et pour lequel les habitants seront 25 fois plus riche au niveau de leur impôt sur le revenu, peuvent très bien avoir la même valeur médiane alors que sur le plan de la richesse de ce territoire, c'est complètement différent, donc ce qu'il faut faire c'est étudier en quartz cette valeur, même si elle n'est pas approprié pour caractériser la la richesse d'un territoire ou du moins sa pauvreté et je pense qu'il faudra vraiment qu'on se penche sur ce problème-là parce que c'est là que la Pierre d'achoppement. Merci monsieur Lamy pour explication de vote. Oui merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, jamais ministre, chers collègues, au je m'exprimerai à la fois sur cet homme dans le monde, dont je fais partie aussi des cosignataires qui a le mérite de poser les problèmes de nos départements ruraux, il existe beaucoup dispositifs depuis, depuis des années, je crois que ça revient, j'ai pris, nous avons pris bonne note aussi de votre engagement, monsieur le Ministre, sur la fiscalité agricole parce que les secteurs agricoles qui les fait vivre ce sont les agriculteurs, malheureusement, on connaît aussi la situation du monde agricole et du monde rural en général et je crois que cet amendement pose aussi le le le problème de l'aménagement du territoire en général et de l'aménagement rural, le management du territoire l'on parle depuis des années, mais sur le terrain réellement qu'est-ce qui se passe de moins en mandat gris culteurs de moins en moins d'activités commerciales, de moins en moins de service public, c'est aussi quand même beaucoup de problèmes Matic et même si on est en loi de finances pour 2018 il y a réellement ce sont les problématiques vraiment du monde rural qu'il faut prendre en compte, il y a des tas de dispositifs qui existent depuis des années, je faisais de la RSR maison le rurales fragiles pour d'excellence le rôle contrat de ruralité, enfin tous les dispositifs, et on sent, on a vraiment de plus en plus de mal de s'y retrouver et je dirais je crois qu'à un moment donné, c'est aussi vraiment un travail de fond qu'il convient d'établir et je pense que là, c'est aussi l'engagement de toutes et tous et donc voilà, c'était un petit peu l'objet de mon intervention, Jean merci. oui, et l'intervention du du rapporteur général du ministre et continue des risques, je le retire.

Collègue donc 538 532 540 ont été défendu le 334 rectifier bis, ce qui a plus. Oui, c'est un amendement complémentaire, je dirais de notre collègue Alain Marquet auquel il tient particulièrement, nous la rappeler régulièrement, on est également dans la dans le classement en ZR des communes membres d'un EPCI à fiscalité propre, l'amendement visant à introduire un critère alternatif à celui de la densité de population secrétaire alternatif serait le déclin significatif de la population depuis les 4 dernières décennies dans les arrondissements à dominante rurale, pourquoi, parce que des communes de toute petite taille, membre d'un EPCI mais dont la densité démographique était levée. Ne peuvent satisfaire la condition d'citer pour être classé en ZR alors qu'elles ont connu un déclin de plus de 30 pourcent de leur population au cours des 40 dernières années, c'est quand même ces communes sont donc désormais rural nous fait nous rappelle qu'un exemple existe en Aveyron, celui de Decazeville auquel il tient particulièrement, qui était autrefois un petit bassin industriel dynamique et qui connaît aujourd'hui de et depuis de nombreuses années de grandes difficultés économiques et sociales, cette petite ville du chef-lieu d'une communauté de communes de 19517 habitants a connu une décroissance de sa population qui est passé de plus de 13000 habitants. Au temps de sa splendeur un peu plus de 5000 habitants, aujourd'hui elle n'est ni éligibles à la DSU. Ni au classement en zone de revitalisation rurale.

Merci, cher collègue, monsieur le rapporteur de l'avis de la Commission sur ces 4 amendements, discussions communautaires. On a à nouveau l'illustration et la réforme de la derrière veut dans la précipitation, sans évaluation sans débat, sans estimation sans simulation est imparfaite, la preuve c'est qu'il y a des amendements sur tous les bancs, visant à réintroduire ensemble de critères qui vise à réformer, encore une fois c'est c'est. Une balle transitoire, je pense qu'il faut se donner le temps de la période transitoire, et d'ailleurs dans le bloc suivant Jorane amendement auquel j'espère le gouvernement sera favorable permettant d'aménager ces bêtes transitoire de nous le temps dans cette trajectoire de revoir et de remettre à plat ce régime de la jet d'erreur parce que il faudrait pas encore une fois prendre ce matin, fin de matinée, des décisions qui conduirait dont on ne mesure pas les effets, je je prends et c'est le cas des amendements qui visent à apprécier les critères au niveau départemental, j'ai aucune idée sur le nombre de communes concernées sur les ailes et les effets que ça peut avoir, c'est la raison pour laquelle la commission émet un avis de retrait demande de retrait sur ces amendements avec une nuance pour le 334 qui vise une situation qui est défendue à l'instant extrêmement particulière parce que les communes en très fort déclin démographique, quand on voit les écarts de 30 pourcent ça doit concerner un nombre extrêmement limité de communes et donc, évidemment, n'est pas dans une suite, il faut une réforme de même ampleur que les amendements, les autres amendements et donc c'est la raison pour laquelle, sur ces 334 c'est une c'est une David sagesse pour le reste demande de retrait sinon avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, la ville du gouvernement. Oui, même chose : avis défavorable aux invitations au retrait, je pense que c'est pas de bonne politique de redéfinir maintenant les critères de définition des adhérer alors même qu'on vient de les changer et de les redéfinir, j'ai bien vu d'amendement spécifiques sur les communes qui aurait perdu 30 pourcent de leurs habitants au cours dernières années ce qui est un chiffre évidemment considérable l'simplement nous n'avons aucune évaluation du nombre de communes concernées, aucune évaluation par conséquent de l'impact sur les finances publiques, donc c'est la raison pour laquelle je confirme un avis défavorable en revanche, certaines propositions d'améliorations qui peuvent être faites par la suite, qui je crois seront faites par le rapporteur général, dont nous discuterons de manière plus ouverte. Merci monsieur le ministre, Monsieur Ruquier les 3 amendements sont retirés ou. Il y a une demande de retrait, mais ils sont maintenus.

Qui s'abstient, il n'est pas adoptée. J'ai même vote pour le 539 même vote pour 540 sur le 334 rectifier bis qui a eu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du gouvernement qui est pour.

Monsieur Jean Sanitas à compter du 1er juillet 2017 a eu pour effet de faire sortir de nombreuses communes du dispositif des RR 100 cas mécanisme de transition ne soit prévu, nous notons que l'amendement à votre initiative, Monsieur le ministre, votée à l'Assemblée nationale à titre provisoire, maintiennent les communes jusqu'au 31 12 20 12 2019 va dans le bon sens l'amendement que nous, nous vous proposons étant jusqu'au 31 décembre 2022 le bénéfice du dispositif des zones de revitalisation rurale aux communes qui en était sorti, le gouvernement a récemment présenté devant le parlement, le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2020, 2 avec pour ambition de construire un cadrage pluriannuel sur cette période d'imposer une trajectoire aux finances publiques en corrélation avec les priorités gouvernementales, dans une logique décentraliser cette ambition devrait être décliné à l'échelle locale une pérennité du dispositif jusqu'au 31 12 2020, offrirait une meilleure visibilité fiscale et financière, tant aux entreprises bénéficiaires qu'aux communes concernées ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie tributaire pour partie de leurs recettes de ce zonage, le gouvernement aura remettre avant le 1er juin 2021 rapport sur la mise en oeuvre de la sortie progressive du dispositif des zones de revitalisation rurale pour les communes concernées qui saura orienter les choix budgétaires à cet horizon. Merci, cher collègue, de 125 rectifier bis qui le défend. Il est fondu. On considère qu'il est défendu.

cette amendement situe dans le prolongement de la conversation qu'on vient d'avoir, il s'agit de donner un peu plus de temps pour faire évoluer les zones de revitalisation rurale et nous proposons de remplacer 2019 à 2020, pourquoi 2020, mais tout simplement parce que ça correspond avec les contrats de ruralité. Merci, monsieur le rapporteur, l'amendement 104 de la commission et puis la vie sur les autres amendements. La l'amendement 104 de la commission et puis qui est aujourd'hui. Je partais à la fois le CIV également voudrait profiter pour vous donner la vie sur les autres amendements qui vient d'être défendu

tous les détenus 30s en 2019 sera le 30 juin 2020, ce qui a l'Avantage d'avoir un délai unique par par la montagne, donc par conséquence je proposerai aux auteurs des amendements, s'ils veulent bien de se rallier à cet amendement, la commission à l'amendement 104 de retirer leurs amendements. Merci, Monsieur le Ministre. Voilà une proposition intelligente, fine cohérente du rapporteur général d'ailleurs, on est samedi, à quelques jours de Noël, on nous fait l'amitié d'être présent, c'est presque l'heure de déjeuner donc bon. Donc, avis favorable sur l'article 104 l'amendement 104 pardon du rapporteur général et les propositions de retrait pour les autres amendements ou avis défavorable d'autres amendements.

Oui c'est amendement a pour but de compléter le rapport parce que effectivement on ne soigne le malade mais on ne s'attaque pas tout à fait à la au mal dont il souffre et donc je reviens sur mon mon prof la problématique du critère de revenu médian qui me paraît totalement inapproprié et il serait utile que dans le rapport qui sera fait, on étudie la pertinence de ce critère pour et je pense très sincèrement que le revenu moyen reflète beaucoup plus le problème des territoires en déserrance alors, simplement, je m'aperçois que l'amendement, elle n'est pas tout à fait bien rédigé donc je préférerais je peux donc le le sous-amendé et on on a dit quand ce rapport étudie la pertinence qu'il y a à substituer aux critères existants, le revenu médian et non pas qu'il y a eu parce que sinon il n'aurait pas toute sa cohérence. Merci l'avis de la commission favorable, Monsieur le Ministre.

excusez-moi je je reprends, si vous le permettez Monsieur Président dans le sous-amendement, je préférerais qu'on indique qu'il y a eu à substituer puisque pour l'instant, le critère du revenu médian s'applique, puisque la loi est applicable et donc ce qu'il faut c'est qu'on vérifie la pertinence qu'il y a eu

Sagesse. Sagesse pour Monsieur le Ministre, donc qui est pour cet amendement 447. Qui Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté. Nous poursuivons avec le l'amendement 105 de la Commission. Rédactionnel favorable, avis savoir Monsieur le Ministre, qui est pour cet amendement. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté, donc je vais suspende la séance, elle sera reprise à 14 heures 30 pour la suite de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2018 nous avons examiné 88 amendements au cours de la matinée, il en reste 293 à examiner la séance est suspendue.